madame la présidente, et je suis sûr que vous approuvez cette mise au point puisque je souhaiterai apporter les rectifications de vote sur les scrutins numéro 117 118 119 et 120 pour lesquels Madame Valérie Létard souhaitaient voter pour un Acte est donné de votre mise au point, cher collègue, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique des scrutins concernés alors nous reprenons la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée visant à protéger les victimes de violences conjugales dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 8 heures et à l'article 8, nous avons, pour commencer, une demande de parole de Madame Michelle Meunier, chers collègues. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, ce chapitre est essentiel dans la lutte contre les violences conjugales et pour la protection des victimes, il s'agit de permettre une meilleure prise en charge judiciaire au travers d'un meilleur signalement des suspicions de violences afin que les agresseurs ne bénéficient pas de plus longue complaisance ce signalement au procureur, qui étaient effectués par les médecins et les professionnels de santé doit être dérogatoire au secret professionnel, ce qui est clarifié ici, c'est que le médecin qui signalent des violences au sein du couple auprès du procureur ne commet pas d'atteinte au secret professionnel habituellement punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, je ne pense pas que cela entache la confiance établie entre la victime qui consultent et le généraliste, je pense au contraire qu'il est urgent de rétablir la hiérarchie des secrets d'un côté, le secret de la violence confiné au sein du foyer familial Un secret destructeur et de l'autre côté, lorsque cette violence est enfin perçu palpable au sein du cabinet médical, ce secret du médecin qui se bornerait à soigner à panser les plaies. Et à ne pas accompagner la victime vers un horizon plus protecteur, ce secret protège l'agresseur lui permet de recommencer à humilier anéantir frappée, violée, il doit s'effacer, plus de lien de confiance entre une patiente et un médecin, mais du lien de confiance entre la victime et le reste de la société, celle qui soigne comme celle qui juge et qui punit protégeons aussi les enfants co-victimes des violences conjugales, cela a été dit tout à l'heure, ils entendent les humiliations se construise durablement dans l'idée que l'un des 2 parents domine l'autre par la coercition la menace, la force, ils assistent aux brutalités il subissent directement parfois ou s'interpose placée dans le rôle de l'arbitre du témoin, les enfants sont les détenteurs d'un secret ils se savent menacés s'il révélait le drame familial, nous devons faire primer la révélation du secret par le médecin ou le professionnel de santé qui ne risque rien pour protéger l'enfant victime car, comme le démontre depuis tant d'années et magistrats, tels Édouard Durand protéger la mer c'est protéger l'enfant.

3 septembre dernier le 1er ministre avec la secrétaire d'État lancé le Grenelle contre violences conjugales, sur la base de ce constat terrible que vous que vous connaissez en 2018 se sont, qui 149 personnes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint 121 femmes également vingt-huit 28 ce constat n'est pas acceptable et ce constat n'est pas une fatalité, c'est tout l'objet de nous ne discussions depuis le début d'après-midi, l'article 8 de cette proposition de loi est issu directement de ces travaux du du Grenelle, travailler en lien étroit avec les associations de victimes et avec les représentants des professionnels de santé, elle vise non pas à lever le secret médical, comme j'ai pu l'entendent comme nous avons pu l'entendre dire, mais à ne pas pénaliser les médecins qui seraient hésitants à faire un signalement au procureur de la république, lorsqu'une vie est en danger, alors, nous entendons naturellement les points de vigilance qui sont exprimés sur ce sujet, ils sont tout à fait légitime au regard des situations de grande souffrance et de détresse que traversent les victimes de violences conjugales, mais qui peut se satisfaire. Qui peut se satisfaire que seulement 5 % des déclarations sont réalisés par des professionnels de santé qui pourtant sont en première ligne pour prendre soin des victimes alors le secret médical et plus largement le secret professionnel n'est pas un sujet évidemment à prendre à la légère, il s'agit du fondement de ce colloque singulier de la relation de confiance d'un d'un patient vers son médecin qui est fondée sur le serment d'Hippocrate, dont vous connaissez les termes admis dans l'intimité des personnes je tairai les secrets qui me sont confiés, reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et c'est la raison pour laquelle ce texte n'altère en rien le secret médical, le code de la santé publique n'est pas modifiée. Le code de déontologie médicale et évidemment préservé et la confiance d'une victime envers son professionnel de santé est ainsi préserver ce qui est proposé avec cet article, c'est de respecter une autre partie du serment d'Hippocrate moins connue peut-être, je vous la cite j'interviendrai pour protéger les personnes si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité. L'article 8 prévoit ainsi sans modifier le secret professionnel, de ne pas sanctionner le professionnel qui fait un signalement au procureur de la République lorsque la vie de la victime est en danger immédiat. Cet article est issue de ses discussions avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment avec l'Ordre des médecins, dans un communiqué du 18 décembre 2019 d'ailleurs, l'Ordre des médecins a soutenu publiquement l'évolution de cet article, devant 226 14 du code pénal, mesdames et messieurs les sénateurs, il s'agit ici d'une disposition qui protège. Qui protège les professionnels de santé qui jusque-là pouvaient hésiter à faire ces signalements. Mais un texte qui protège également évidemment surtout les victimes de ces violences conjugales pour éviter le scénario, les scénarios du pire voilà Mesdames et messieurs les sénateurs, ce qui fondera pour la suite, nos avis défavorable sur les amendements de de suppression et qui guidera nos prises de position sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Très bien, merci, monsieur le ministre, je donne maintenant la parole à Madame Benbassa pour défendre l'amendement 13 rectifié. Seul président. Merci madame la présidente, monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nul ne peut nier et l'effet délétère de l'plus psychologique dans un couple notamment lorsque celle-ci est nourrie par la peur et les pressions morales pour de nombreuses victimes de violences conjugales, la première étape est celle du délit, une personne battue par le conjoint ou compagnon dont elle est amoureuse refusent souvent de se considérer comme une victime, elle finit d'ailleurs bien souvent estimait responsable des attitudes violentes de son compagnon à son égard se rendent cependant parfois dans les hôpitaux afin de faire constater et soigner leurs blessures, nous ne souhaitons pas comme le préconise l'article 8 que le médecin soit autorisé à donne lancer les actes de violence qu'il a pu constater sur sa patiente auprès du procureur de la République nous estimons en effet qu'une telle atteinte au secret médical pourrait se révéler contreproductive et pousser les victimes de violences conjugales à renoncer aux soins médicaux, il est impératif que le lien de confiance existant entre les patients et le personnel soignant soit maintenu ainsi a-t-il proposé par le présent amendement de supprimer l'article 8 merci. Merci madame Benbassa. ça donne la parole à Madame, la rapporteure pour l'avis de la commission. Merci madame la présidente, ma chère collègue donc vous proposez de supprimer l'article 8 comme monsieur le ministre a expliqué tout à l'heure le serment d'Hippocrate, c'est quelque chose de très particulier quand on prête serment d'abord, on vous donne une sorte de toge, moi je me souviens d'été ça avait marqué parce qu'il a été usé crasseuse, c'est-à-dire que pour moi il y avait beaucoup de de père de confrères qui m'avait précédée et quand on prête serment ça veut vraiment dire quelque chose, mes yeux ne verront que ce qu'doivent voir et ça reste un secret, c'est un secret partagé qui protège le patient qui n'est pas là pour protéger le médecin mais pour protéger le patient et garder ce lien un peu mystérieux qui se tisse au fil des consultations au fil des années et qui permet de respecter la parole qui est donné, quand on a relu cet article 8 avec cette proposition je crois que c'est vraiment contraire à la vie de la position que de le supprimer, parce qu'en fait, nous l'avons améliorée pour faire en sorte que nous maintenions ce secret entre le patient et le médecin, c'est vraiment une protection, une garantie donc je je crois que c'est admis qu'on puisse déroger au secret médical, c'est prévu par la loi compte cette obligatoire pour la survie de notre patient, bien évidemment, ça ne nous pose pas de questions, mais je pense que cette crainte que vous exposez n'est pas justifié et que cet amendement n'a, n'a pas sens parce qu'il n'ait n'élargit pas considérablement le Champ du secret, donc je vous proposerai de

je veux, il n'y a pas de demande d'explication de vote je mets donc aux voix l'amendement 13 rectifié, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous passons à l'amendement 14 rectifier, il est toujours présenté par Madame Benbassa. Merci monsieur le président, madame la rapporteure, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, comme nous avons pu le dire précédemment, l'article 8 autorise le médecin qui a constaté des marques de violence sur le corps de sa patiente a dénoncé la situation auprès du procureur de la République, une telle proposition contreviendrait de manière évidente au secret médical, celui-ci constitue pour les patientes et patients, une garantie de liberté d'échange avec les représentants du corps médical, il favorise l'instauration d'une relation de confiance indispensable au bon déroulement des soins et du traitement, il n'est de ce fait aucunement souhaitable que le médecin se transforme en un rouage de la procédure judiciaire à la presse à la place du rôle des dénonciateurs que l'article 8, souhaite, lui, a signé, nous préférons que le personnel hospitalier est un devoir de conseil et d'accompagnement envers la victime, nous considérons donc par le présent amendement qu'il pourrait être pertinent que le personnel soignant puissent diriger les patientes ayant subi des sévices au sein de leur foyer vers des associations en charge de lutter contre ces violences, celles-ci sont en effet les mieux armés pour rassurer les victimes leur apporter un soutien moral, les éclairer sur leurs droits et 20 éventuellement les accompagner dans le cadre des procédures judiciaires qu'elle souhaiterait entreprendre la mesure que nous proposons est donc une alternative à la fin du secret médical pour les victimes de violences conjugales que comporte l'article 8 je vous remercie. Merci madame la présidente, donc bien sûr un médecin pourra toujours orienté vers une association vers une structure de prise en charge adaptée et souvent nous le faisons et et je voudrais remercier et féliciter les associations qui prennent en charge et des victimes, qui font un travail extraordinaire, mais malheureusement cet accompagnement social de la victime n'est pas toujours suffisant, donc il ne faut pas vraiment se savoir prévenir la justice qui souvent a les moyens de mettre un coup d'arrêt à la violence du du conjoint c'est stopper l'agresseur, qui doit être notre but et je crois que vraiment il faut conserver l'article 8, telle que nous l'avons amendé et non pas de réécrire complètement, donc c'est un avis défavorable.

je, je regrette que les les 2 amendements que nous savons, Esther Benbassa a a présenté et qui sont donc co-signé par l'ensemble du groupe ne fassent pas plus débat. Parce que, outre les problèmes qu'elle a tout à fait pointer il y a aussi une certaine réaction de beaucoup d'associations féministes notamment qui pointe un certain nombre de contradictions et j'ai entendu effectivement madame la secrétaire d'État, je crois que c'était à l'Assemblée nationale qui a aussi montré des contradictions, c'est-à-dire qu'à la fois on est tous et toutes, conscient du phénomène de l'emprise que subit une femme donc sa paralysie parfois à pouvoir exprimer et et dénoncer les violences tout l'importance d'être soutenus, accompagnés par des professionnels de santé qui vont l'aider à cette prise de conscience, mais on sait que par compte combien, comment elle va faire pour réagir et à ce qu'elle va le faire rapidement ou pas, ça c'est un un autre problème, donc il y a cette contradiction-là

d'emprise comme des être mineure qui ne serait pas en capacité. De, de, de faire les choix qu'elles ont assumé, c'est-à-dire elle-même de se prendre en main et de dire oui effectivement, grâce à l'accompagnement du du des, des personnels de santé, je vais porter plainte etc donc, d'où le le l'amendement qui a été présenté en 1er de suppression de l'article 8 parce que l'article 8 n'est pas du tout nuancé même si la commission n'a amélioré un certain nombre de contours, je le concède, tout à fait et j'en remercie Madame la rapporteure et la 2ème chose compte Esther Benbassa dit que ça serait quand même important de notifier que le médecin le professionnel puisse donner les coordonnées les adresses des associations féministes les réponses de Madame la rapporteure sont insuffisantes quand elle dit : mais non, ça doit être la justice, bien sûr, ça doit être la justice, bien sûr, ça doit être la police mais il faut aussi qu'il y a un accompagnement psychologique, un accompagnement de soutien qui est opéré par les associations. Qui ont besoin d'ailleurs de moyens financiers, de moyens humains, pas seulement d'être salué quand ça nous arrange. Effectivement, j'ai entendu comme vous quelques associations féministes qui déplorait le fait que cet cet article viserait à considérer, je mets beaucoup de guillemets, je résume les femmes comme étant en incapacité donc certaines disait ça voudrait dire que les femmes seraient comme des mineurs et qu'elle ne pourrait pas prendre leurs propres décisions pour elle-même et philosophiquement c'est très dérangeant. Je crois que ce débat s'entend, et la question peut se poser, vous avez tout à fait raison de le soulever, néanmoins, je pense que quand on parle là de situations d'urgence et de situations de vie qui doivent être sauvés, on ne peut pas dans le même temps, dire que notre mot d'ordre à tous et ne rien laisser passer, c'est faire des campagnes pour que les témoins interviennent dans les violences contre les femmes, mais aussi dans les violences en direction des enfants et dire que c'est l'affaire de toute la société qu'on ne doit pas fermer les yeux et et en même temps, risquer de voir parfois des médecins ou des soignants être parfois sanctionnés parce que c'est ce que certains nous ont dit parce qu'ils ont souhaité alerter sur cette question des violences conjugales, donc je crois que c'est extrêmement important de pouvoir permettre cela, et faire en sorte que les médecins qui ont face à eux des femmes qui ne sont pas tout à fait décidés à alerter elle-même les forces de l'ordre puissent le faire, et puis je voudrais dire, et on sait très bien, puisque ici nous sommes au sénat dont chacune et chacun d'entre vous le sait, on n'est pas dans des situations qui sont forcément toujours comme on les imagine dans la théorie, et il arrive, c'est une réalité, c'est difficile, temps mais vous le savez, c'est la réalité, parfois il y a des femmes qui refusent de porter plainte, qui refuse que qu'on appelle à l'aide qui refuse qu'on intervienne alors qu'elles-mêmes sont en danger de mort et je crois que dans ces cas-là, oui, il est important qu'une autre personne puisse intervenir et enfin puisque vous évoquez la la question des moyens, je voudrais rappeler que nous avons ouvert pendant le confinement en fonds exceptionnel d'un montant de 1 1000000 d'euros, pour soutenir les associations locales de terrain et je voudrais dire que ce fonds n'est pas entièrement utilisé et que donc ce fonds est toujours ouvert et je le redis, je le redis, sans cesse, si vous avez connaissance d'associations locales de terrain qui sont en difficulté ou qui, par de nouveaux projets et qui ont besoin de davantage de subventions, nous avons dégagé les moyens pour cela et donc il faut absolument qu'elle puisse faire remonter au service des droits des femmes, leurs dossiers de subvention pour qu'on puisse attribuer concrètement cette somme que nous avons dégagé pendant le confinement, je vous remercie. Merci madame la ministre madame de La Gontrie, vous avez la parole pour explication de vote. Merci madame la présidente, je regrette que l'amendement qui est présenté à l'instant, ne soit pas un amendement de complément parce que la proposition qui est faite est évidemment pertinente mais je rebondirai sur. Ce qui a évoqué notre collègue Laurence Cohen, elle a raison, nous aurions dû débuter par un débat, c'est-à-dire comment concevons-nous entre nous parce qu'ensuite les amendements ne sont que la mise en oeuvre de ce que nous allons, considéré comme le plus pertinent, le débat, il est de savoir si premièrement nous considérons qu'il faut à chaque fois que cela est possible, dénoncer les faits de violence conjugale et donc les faits de violence subies par une femme, point numéro 1. Il n'est pas exact de penser qu'il n'y a que le médecin qui peut le faire, chacun de nous peut le faire, donc il n'est pas exact de penser que seul un médecin peut venir en aide la 2ème chose c'est qu'en est-il de du rapport entre le médecin et sa patiente à quel moment est-ce qu'il est le plus efficace. De déclarer des faits à la justice, est ce que c'est au médecin de le faire, ça c'est la bonne question et pour ma part, je ne suis pas médecin, j'ai essayé de comprendre et d'entendre les médecins qui pratiquent beaucoup ce genre de question. Et pour une bonne part, certains disent attention si la patiente n'a plus confiance dans le secret de notre cabinet. Elle pourrait dans ce cas-là, ne plus s'y présenter, c'est une question légitime, d'autres y compris au sein de notre groupe, disent, peu importe, allons-y, il faut signaler, moi j'ai tendance à penser personnellement et nous sommes un certain nombre dans mon groupe à avoir signé un amendement qui prévoit qu'il faut l'accord de la patiente, ce qui est très intéressant, c'est ce qui a été le débat qui a été entamé entre Laurence Cohen et et la ministre Chiappa il faut savoir que le secret professionnel, on peut y déroger que dans un cas où effectivement ce sont des violences ou des maltraitances mais avec l'accord de la victime 226 14 du code pénal, le seul cas où le corps de la victime n'ait pas demandé, c'est lorsqu'il est mineur, donc on est exactement dans cette situation, on considère donc je ne dis pas qu'on a raison ou tort mais je précise des choses, on considère donc que le fait d'être sous emprise. Revient à être mineur. Et là, c'est une question importante, parce que pour ma part, je pense que être sous emprise, bien sûr, ça nécessite un accompagnement particulier, le médecin est là pour ça, est ce que pour autant, considère que c'est un mineur non et donc c'est pour cela que pour ma part avec un certain nombre de collègues, j'ai proposé un amendement qui valide l'intégralité du dispositif qui est proposé, qui a le mérite d'ailleurs de citer, pour la première fois dans le code, le mot emprise mais qui demande que la patiente et donné son accord, autrement nous allons détruire le lien de confiance qui est utile, évidemment, dans cette séquence entre le médecin et sa patiente. Merci, cher collègue, s'il n'y a plus de demandes d'explications de vote, je mets aux voix l'amendement 14 rectifié, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui compte. Alors on recommence parce que vous vous levez-vous : baissez vos mains, donc on va recommencer, qui est pour. le 14 rectifié qui est. Pour qui est contre. Qui s'abstient l'amendement n'est pas adopté alors, nous passons à l'amendement numéro 49, il est présenté par Madame Menier. Merci madame la présidente, cet amendement vise à préciser explicitement dans la loi, l'obligation de signalement par les médecins de suspicion de violences sur mineur, je rappelle que cet amendement a été adopté par le Sénat en juillet 2018 lors de l'examen de la loi de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, il n'avait pas en revanche passer le cap de la CMP, donc nous avons aujourd'hui l'occasion de rattraper le temps perdu, agents de Les agents de l'État ou de la fonction publique territoriale l'les médecins sont face à un dilemme éthique, soit il est signale ces violences et risquent des poursuites des sanctions disciplinaires des poursuites pénales au regard de la levée de leur secret professionnel après avoir appliqué l'article 226 tiré 14 du code pénal comme ça vient d'être dit ceci allant pourtant à l'encontre des recommandant de recommandations de la Haute autorité de santé soit les médecins donc, où les professionnels de santé ne signale pas et risque d'être l'objet de poursuites et sanctions pénales pour entrave à la saisine de la justice, c'est peut-être ce dilemme qui explique le faible taux de signalement, lorsqu'un médecin détecte des signaux d'alerte qui lui permettent de suspecter des violences psychologiques, physiques ou sexuelles commises à l'encontre de mineurs, l'introduction de l'obligation de signaler par cet amendement permettrait donc de multiplier les taux de cas confirmés de signalement de réduire le risque pour un enfant de mourir des coups qui lui sont infligées permet aussi, donc, cet amendement de réduire un long parcours de souffrance des victimes car le signalement, je le rappelle, est la clé du parcours de soin et ça permet aussi de rompre le cycle de la violence, le plus tôt possible pour prendre en compte en en charge les agresseurs afin que ceux-ci ne récidivent pas plus auprès d'autres mineurs éventuellement. cet amendement, ma chère collègue propose d'instaurer une véritable obligation de signalement à la charge des professionnels de santé lorsqu'ils suspectent qu'un mineur est victime de violences, donc nous avons beaucoup travaillé ensemble, ma chère collègue sur ce sujet puisque nous avions une mission présidée par Catherine Deroche, avec Maryse Carrère et et donc vous-même et nous étions arrivés à la conclusion que l'équilibre actuel, donc qui repose sur une option de conscience qui laisse aux professionnels de santé, la faculté de signaler était satisfaisant, instaurer une obligation de signalement ne mettrait pas fin au dilemme éthique qui se pose à tout médecin qui suspecte, sans en être certain que des violences sont commises sur un mineur, il faut bien comprendre que le médecin est toujours dans un conflit de devoir je signale ou je ne signale pas je protège du mieux possible dans quelle, de quelle façon, c'est ça l'essence même le le vrai souci c'est ce conflit de voir, donc, c'est vrai, ma chère collègue ma chère Michèle Meunier vous avez déjà défendu cette position au sein de notre cours de travail, donc vous êtes vous êtes constante, je trouve ça très bien parce que vous avez votre ligne de conduite, je vous dirais que nous avons la nôtre et que quand nous avions rendu les les conclusions de cette mission de, finalement, nous avons dit que finalement l'équilibre, il était là et qu'il ne fallait pas y toucher, donc je vous propose de rester sur cette mission que nous avions et d'émettre, donc un avis défavorable, mais je vous félicite de garder vos valeurs et votre constat. Madame la la présidente, que ça soit l'occasion pour moi d'abord de saluer à mon tour le travail que vous avez menée avec la sénatrice des rochers avec même la la rapporteure, nous avons eu l'occasion de nombreuses reprises de converser au sujet de votre mission et d'échanger sur la meilleure façon de protéger les enfants contre les violences. L'objectif que poursuit que vous poursuivez avec cet amendement, madame la sénatrice, qui vise à instaurer cette obligation de signalement des violences exercées à l'an compte des mineurs est déjà satisfait en en réalité, je pense que l'introduction cet amendement pourrait créer de la confusion et nous serons d'accord pour nous dire qu'il ne peut y avoir de confusion en ces matières, en vertu de l'article 434 tiré 3 du code pénal, révélé des maltraitances commises au préjudice de mineurs est une obligation légale. 26 tiré 14 ce même code pénal telle qu'il est rédigé délivrent les professionnels du secret médical en cas de privations et de sévices sur les mineurs victimes. En revanche. Il est vrai. Les médecins libéraux signal très peu les violences sur mineur. Seuls 5 à 6 % des signalements sont issus de médecins qui pourtant voit passer tous les jours nos enfants. Alors c'est un des sujets que nous avons décidé d'aborder traité dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants que j'ai présenté le 20 novembre dernier à l'occasion du 30ème anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant,

Vous êtes médecin libéral dans une petite commune, vous êtes le médecin de famille et puis des générations. Vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec ce genre de situation, vous vous sentez seul il y a besoin qui liait. Service ressources une personne ressource qui puisse vous accompagner. face à ces situations, vers lesquels vous pouvez éventuellement renvoyer ces situations-là, c'est ce qui s'est passé dans les faits, et vous, vous êtes très bien placés pour le savoir, madame la sénatrice à Nantes par exemple, au CHU de Nantes, avec le Docteur Fabre qui dé facto depuis 15 ans, 20 ans, ce sont devenus des personnes ressources pour les médecins du territoire qui spontanément, naturellement, se retourne vers et au sein de l'unité d'accueil pédiatrique Enfance en danger pour avoir ce soutien n'est plus être isolé face à cette situation, le plan que j'ai présenté en novembre dernier, prévoit que d'ici à 2022 dans chacun des territoires, nous puissions pourrait du 22 le temps de le déployer se dépêche d'ici 2022, madame, d'ici 2022 d'ici 2020 et le plus vite possible parce que je pense que c'est une des mesures fondamentales, voilà donc les dispositions du texte, elles sont actuellement nous semble satisfaisante. Pas créer de confusion en les modifiant, je l'ai dit et répété, c'est fait l'objet de concertation avec les professionnels de santé, nous avons obtenu un équilibre qui satisfait à à tout le monde et donc je propose un avis défavorable, puisque c'était la question qui m'a été posée initialement. Si Monsieur le ministre, il ne s'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 49 avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

L'amendement n'est pas adopté. Face à la présentation de l'amendement 48 et c'est toujours Madame Meunier. Oui merci, donc cet amendement 48 propose de remplacer les mots estime en conscience par le le mot suspecte alors je résume un peu les épisodes précédents : le texte issu de l'Assemblée nationale, mentionnait lorsqu'il lui apparaît que ces violences en parlant du médecin et en commission des lois du Sénat, je pense que une autre rédaction a été retenu, c'est lorsque le médecin ou professionnels de santé estime en conscience que les violences mettent en danger personnellement donc je je préfère le terme suspecte le médecin ou le professionnel n'a pas à convoquer sa conscience, cet aspect-là, l'option de conscience relève de la doctrine déontologique des soignants et les soignantes reprise dans la partie réglementaire du code de la santé publique, le médecin, je cite, alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, donc c'est le R 4 42 17 tiré 44 du code de la santé publique, il n'y a pas donc lieu de procéder à ce rappel redondant, à mon sens, dans le code pénal, de plus, la consultation ne place pas les médecins ou les professionnels de santé à la place du témoin, ils ne peuvent donc pas, à part leur apparaître des violences ni leurs conséquences, en revanche, ces professionnels de santé sont formés à détecter des signaux d'alerte à l'à repérer des situations à discuter et à interroger les victimes potentielles. Ces médecins ou ces professionnels de santé ne peuvent donc que suspectées d'effets dont les conséquences potentiellement graves nécessitent le signalement pour protéger les médecins en les encourageant à signaler des poursuites ont déjà été engagées à l'encontre de professionnels qui avait signalé sur la base de suspicion de violences exercées par le conjoint après l'examen d'un enfant, conduit par un parent ce signalement se conçoit et doit être favorisé au procureur, ensuite, de diligenter une enquête contradictoire, donc voici qu'exprimer cet amendement. Chers collègues Madame la rapporteure, avis de la commission. donc c'est moi qui ai proposé la Commission la formulation. Estimant en conscience pour bien marquer la responsabilité qui incombe aux professionnels et pour insister sur l'option de conscience qui s'applique en pareille circonstance, option de conscience, n'oubliez pas que le secret professionnel, on ne doit pas y déroger, c'est un secret : quand on est dépositaire, mais il y a pas d'opposition entre nos 2 rédactions puisque votre amendement me donne bien l'occasion de préciser que l'on n'attend pas du professionnel qu'il ait la certitude que des violences sont commises pour pouvoir signaler c'est l'enquête qui permettra d'apprécier ce qu'il en est véritablement je préfère donc vraiment, vous savez la rédaction que nous avons adopté en commission, car elle met bien en lumière le cas de conscience qui se pose aux médecins qui envisage de transgresser ce secret professionnel parce qu'il a acquis la conviction que sa patiente est en danger. Madame la rapporteure, monsieur le ministre pour l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente. La décision de déroger au secret médical, la la rapporteure, a dit constitue une une décision est évidemment éminemment lourde qui doit être prise après une réflexion du médecin et réflexions qui conclut à l'impératif de venir en aide à une personne dont la vie est est en danger, et là on est vraiment au coeur de cette cette tension éthique entre le respect du secret professionnel, d'une part et la réclame la déclaration auprès du procureur d'une situation dont on estime. Elle peut mettre en danger la vie d'une d'une personne. Et cette rédaction d'une estimation en conscience nous semble bien traduire cette position et cette tension éthique de façon équilibrée, contrairement à cette notion de suspecte que vous proposez, qui en réalité relativement neutre, voilà donc pour l'ensemble de ces, de ces raisons, la rédaction actuelle nous nous satisfait, nous paraît équilibré la vie sera donc défavorable sur l'amendement madame la sénatrice. Merci monsieur le ministre, s'il n'y a pas de demandes d'explications de vote, je mets aux voix l'amendement 48 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous passons à l'amendement 11 rectifié c'est madame veut rien qu'il présente. Sa rédaction actuelle prévoit que la dérogation au secret médical peut se faire lorsque ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat. Or, l'utilisation de la terminologie danger immédiat, renvoie à un risque de mort imminente pour la victime de violences, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe en règle générale, dans les violences conjugales et justement on parlait d'emprise et c'est plutôt une mort lente qui intervient, et donc le médecin n'intervient pas au moment du danger immédiat dans ces cas-là, c'est souvent trop tard et c'est plutôt aux urgences, comme je le disais en préambule de de l'examen de cette loi, cette proposition de loi. C'est donc au moment où on pense que la victime est sous emprise, qu'elle n'a pas les moyens effectivement de se défendre tout seul que il faut que le médecin à ce moment-là la compagne et signale et nous sommes bien d'accord, c'est pas le c'est le pas le médecin qui dira : il y a, où il n'y a pas, ce sera ensuite la justice qui aura à faire son travail, mais il est mieux de pouvoir avoir le temps de l'enquête est signalé dès que le médecin a l'intime conscience d'un danger, sans pour autant que ce danger souhaite immédiat.

le secret médical, c'est une garantie essentielle pour les patients mission si on affaiblit ce secret, on court le risque que les patients réellement ne consultent plus leur médecin filles de ne plus confier ou que, même si le médecin devine qu'il se passe quelque chose, on ne revoit plus patient, parce qu'on on est allé un peu trop loin, que ce n'était pas le moment qu'on n'a pas trouvé les bons mots et que la patiente s'est dit je suis découverte, je suis aussi un peu honteuse de voir que je suis battu, ça, ça peut se voir, je l'ai vu et vous ne revoyez puis la passion parce que vous avez deviné, il faut aussi respecter ça et attendre un petit peu, c'est la raison pour laquelle je suis défavorable à l'élargissement proposé par cet amendement, s'agissant de 2 personnes majeures la dérogation au secret médical ne peut être admise que pour sauver un patient dont la vie est directement menacée et ça c'est déjà le cas, le médecin bien sûr peut accompagner la patiente il peut l'encourager à porter plainte, bien sûr, mais il n'a pas vocation à se substituer à cette patiente, sauf en cas de péril immédiat mais ça, on a vu que c'était je dirais par un autre, a-t-il donc le le lien de confiance entre les patients et les médecins, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qu'il faut entretenir faut garder cette confiance et il faut qu'on garde nos nos patientes pour les sauver, plus tard peut-être. Merci madame la rapporteure. Monsieur le ministre à vie du gouvernement. Et ce sera un avis aussi défavorable, madame la la présidente, madame la sénatrice. Simplement précisé qu'il n'y a pas de de risques tels que vous le craignez que les situations dérogation au secret professionnel, soit trop restreinte parce que c'est un peu le sens de de de l'amendement que vous que vous portez ce terme immédiat il porte bien sur le, sur le danger, non pas sur le sur possibilité de dérogation au secret médical va donc bien au-dessus de la des seule situation où il existe un risque vital immédiat et madame la rapporteure, là c'est bien précisé, voilà, il nous sommes importants par ailleurs même de caractériser et de qualifier le risque qui pèse sur la victime avec cet cet adjectif, une fois encore, c'est aussi la formulation qui a obtenu une forme de d'équipes de consensus avec l'Ordre national des des médecins, voilà donc pour l'ensemble de ces raisons, ce sera un avis défavorable. Merci monsieur le ministre madame de La Gontrie, vous avez la parole pour explication de vote. Merci madame la présidente. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, notre collègue rapporteur. Et j'ai trouvé qu'elle plaidait formidablement bien, pour que l'accord de la patiente soit une condition indispensable. à ce dispositif. En expliquant sa qualité de médecin, ce que je n'ai jamais été à quel point il était important de préserver. La qualité de cette relation et comment est-ce que pour des, des, des, des patients ne pouvait être évincé de cabinets médicaux si justement le risque de non-respect du secret était trop grand, parce que l'amendement qui est proposé par notre collègue rien effectivement élargi. Le nombre, enfin le le le Champ dans lequel il serait possible de ne pas respecter le secret. la vie, la, la victime, la patiente ne seraient pas d'accord. Donc. Personnellement, je ne peux pas partager ce point de vue puisque je demande qu'il y a l'accord de la patiente. Et lorsque j'entends la rapporteure soutenir qu'effectivement. La patiente sous son point de vue le fait qu'elle continue de revenir dans ce cabinet, parce qu'elle aura confiance est important. Plaide à la fois pour l'amendement que j'ai présenté après pour maintenir l'accord de la patiente, et effectivement, elle en compte de ce que vous proposez et moi en cohérence, parce que je veux l'accord de la patiente et j'ai vu un cas très restreint de non respect du secret médical, je ne souhaite pas soutenir cet amendement. Merci, cher collègue, alors Madame rien pour explication de vote. Je vais malgré tout essayer de, de, d'expliquer, lorsqu'on est sous emprise, on n'a pas le moyen de se défendre seul et si on n'est pas aidé et accompagné on ne on n'y arrivera pas, et le médecin fait partie de ceux qui peuvent aider ou accompagné maintenant

donc je je vais retirer mon amendement, mais clairement l'emprise est quelque chose qui fait qu'on ne peut pas demander à la personne sous emprise de d'avoir une décision éclairée. Pour soi-même. Merci, cher collègue, et donc si j'ai bien compris la maman 11 rectifié et retiré, nous passons donc à l'examen de l'amendement 21 rectifié bis présenté par Madame de La Gontrie. Merci madame la présidente, pour que les choses soient claires aujourd'hui, il est donc dit que le médecin doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure s'efforcer de. Mais s'il ne l'obtient pas, il peut quand même faire le signalement. S'efforcer de d'une formule qui a sans doute été introduite pour dire qu'il était quand même prié d'essayer de convaincre et c'est une bonne chose mais. Il peut donc s'en passer, sachant que, il faut tout à la fois la situation danger immédiat et la situation d'emprise, donc j'ai largement déjà développé les motifs pour lesquels il semblait un grand nombre de praticiens qu'il était important de maintenir la relation de confiance et donc de secret entre le patient et son médecin et c'est pour cela qu'il est proposé de supprimer ce membre de phrase qui disait en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il faut que le médecin, et cet accord pour pouvoir signaler. oui ma chère collègue, donc j'étais parfaitement d'accord avec avec votre introduction, mais la fin de la phrase était vide. Sauf en cas de danger immédiat et en prise alors l'emprise qu'est ce que c'est l'emprise c'est une prise de possession du psychisme de l'autre, c'est difficile de s'en rende vraiment compte l'emprise, c'est comme un vampire qui vient aspirer votre volonté, vous n'avez plus de volonté quand vous êtes sous emprise vous subissez en permanence une influence abusive une affluence possessif négative, c'est ça, l'emprise l'emprise, c'est quelque chose dont on ne peut plus se dégager, puisqu'on est sous emprise, on ne s'en rendent même plus compte on est poussé, on n'a plus son propre c'est psychisme est tellement que compte le bourreau, je vais l'appeler comme ça, pour mieux expliquer quand le bourreau n'est pas là la victime, elle est quand même sous emprise et s'il lui dit : tu n'es qu'un déchet quand je ne serai pas là tu mangeras tes déchets, elle le fera, même s'il n'est plus là, parce qu'on ne s'appartient plus quand on est sous emprise, on est dépossédé d'une partie de soi-même. C'est quelque chose de mystérieux, effectivement, il faut s'en libérer, c'est très spécial et il faut diagnostiquer la patiente sous emprise donc à la fois le danger immédiat et l'emprise et là il faut aider cette patiente, bien sûr, elle n'existe plus, par elle-même, vraiment, elle n'existe plus, c'est très intéressant de comprendre aussi comment l'emprise s'installe avec d'abord une phase de séduction puis la plus belle ensuite de dénigrement, tu es la plus moche et puis après. c'est normal que je voilà, parce que je ne veux rien, je ne suis rien etc etc et c'est : c'est la piste qui qui qui, voilà qui va vers les bas-fonds chacun abrite à l'intérieur de soi-même, c'est très compliqué et il faut le diagnostiquer, parce qu'il faut sauver ces patientes, elles ont besoin d'aides, elles sont besoin d'une thérapie, donc vraiment je j'aurais 10 mots d'équilibre qui était dans dans la rédaction de l'article 8 avec la personne en de immédiate et en prise et là, avoir l'accord de la victime, on ne leur a jamais les sous emprise et pourra pas donné son accord. Merci madame la rapporteure avis du Gouvernement Monsieur le Ministre. Merci madame la la présidente tandis que cet amendement supprime la possibilité de dérogation au secret professionnel, qui est l'avancée qui est au coeur de cette article avis sera défavorable Mais que ça soit l'occasion pour moi aussi. Et de rappeler que les dérogations au secret médical existe déjà, notamment pour les mineurs et les personnes vulnérables et d'ailleurs, dans le droit actuel. C'était en renvoyant les femmes aux personnes vulnérables que des dérogations pourraient être prises, et c'est la raison pour laquelle ce texte prévoit une 3ème voie pour que justement demain nous ne renvoyons plus les femmes à un statut de mineur de personne vulnérable, contrairement à ce que vous évoquiez les unes et les autres, tout à l'heure. 3ème voie qui a été, je le redis, établi avec l'Ordre national des médecins et qui, une fois encore, permet à la fois garder la confiance de la personne envers son médecin tout en donnant cette protection supplémentaire pour les victimes de violences absolument nécessaire. Moi je pense qu'il faut quand même rester, comment dirais-je, équilibré dans dans la façon dont on présente les choses, l'emprise, ça n'est pas quelque chose de démoniaque, comme dans un film d'épouvante et c'est effectivement le fait que petit à petit. Le le le bourreau. Va instaurer. une relation qui va dévaloriser la personne avec qui il se trouve et d'ailleurs pour qu'il y ait, violence physique, mes chers collègues, pour qu'une une femme parce que c'est une majorité de femmes se laisse frapper ne ne réagissent pas, c'est qu'elle est déjà sous emprise psychologique, c'est-à-dire à l'été, dévalorisé dévalorisé dévalorisé, ce qui fait qu'elle va, elle va penser que finalement elle le mérite bien après il y a des tas de mécanismes quand je dis raison garder, c'est parce que quand Mes chers collègues, certains d'entre nous, peut-être que ça m'arrive, défendons tels ou tels amendements, on va se laisser emporter par cette, cette espèce de passion, je suis quand même très étonné parce que si l'emprise. Et telle que ça a été décrit et je le partage, c'est un phénomène que je partage avec les nuances que j'ai apporté, je ne comprends pas pourquoi vous avez rejeté l'amendement 14 ma collègue, Esther Benbassa, qui demandait simplement à ce que dans la loi, figure le fait que le médecin puisse signaler à la patiente la la possibilité de se de contacter des associations pour l'aider pour l'accompagner donc il y a quand même quelques petites contradictions vous acceptez des choses madame la rapporteure quand tout ça va dans le sens de ce que porte la commission et puis finalement sur d'autres amendements, c'est un petit peu différent, donc c'est pour ça que je, je, je vous appelle parce que je sais que vous avez l'esprit de justice a un peu d'équité et ça c'est la première, la première chose que je je veux donner et nous voterons. L'amendement qui est, qui est présenté, par ma ma collègue parce que, effectivement, il a les nuances qu'elle a fort habilement présenté et donc c'est pour ces raisons que nous allons voter pour. Madame Cohen, Merci madame la présidente, et je voudrais faire un petit point en psychanalyse, l'emprise n'est pas diaboliques, c'est une relation perverse de soustraire avant de diriger la personne a porté plainte, il faudrait surtout qu'il s'en rendent compte qu'il y a en prison et qu'il faut soustraire. La personne violentée de cette emprise donc il y a un vrai travail à faire pour le médecin, et parfois les coups ne se voit pas, et puis il ne faut pas décrire l'emprise de cette façon-là, excusez-moi, il peut y avoir une emprise sur son employé sur ses enfants sur le voisin enfin l'emprise et diverses et je crois que il faut admettre que la perversité tellement complexe que l'emprise est tout aussi complexe, alors vraiment c'est une relation très difficile à dénouer et que si elle n'est pas dénoué : vous pouvez envoyer le conjoint, là où vous voulez le l'accompagner, lui, de je sais pas Lucie lui faire faire un stage, ça ne servira à rien parce que les pervers ne guérissent pas en plus Merci madame la présidente, je vais également voté cet amendement parce que je pense qu'il est mesuré par rapport au précédent amendement et en réalité, on vous l'avez dit vous-même dans l'exposé tout à l'heure des faits, très peu de signalements de la part des médecins, on doit s'en étonner, et on doit aussi peut-être mettre en place des mécanismes qui vont faire que les médecins vont être poussé un peu plus incités à se à signaler et donc cet amendement je pense les y incite et préserve malgré tout le le secret médical, puisqu'ils le feront, à condition que la victime soit d'accord, donc bien entendu, je voterai cet amendement, je vous remercie. Merci, cher collègue, il n'y a plus de demandes d'explications de vote, je vais donc mettre aux voix l'amendement 21 rectifié bis qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

On recommence, qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté. Alors l'amendement 50 présenté par Madame Menier. Menier. Sa présidente, cet amendement, été le corollaire de la l'amendement 48 sur l'obligation de signalement puisque il a été rejeté en cohérence, je retire l'homme non, devant 50 mais Madame la rapporteure a raison, je suis tenace, donc je reviendrai. Merci madame Meunier, l'amendement 50 et donc retiré je mets aux voix, l'article 8 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, l'article 8 et adopté alors article additionnel après l'article 8 un amendement 80 il est présenté par Madame Cohen. Oui, ils complètent, finalement les amendements que nous avons déjà présenté, même s'ils avaient été rejetés et puis il contribue encore à enrichir notre notre discussion parce que nous pensons effectivement que si il y a un pas l'accord de de la victime, le signalement, donc peut être tout de même fait par le le médecin, c'est ce qui a été voté majoritairement dès lors que la victime en est informé, donc c'est pas seulement l'accord de la victime, c'est son information qui prévaut, donc effectivement là on peut se dire que, il y a besoin dans ce qu'elle a de garantir la mise en sécurité de la personne qui est visé par un tels signalements contre le fait qu'elle est réellement consentis et nous proposons dans ces cas-là, que le juge aux affaires familiales puisse délivrer en urgence une ordonnance de protection pour ces victimes, comme le souligne Gilles Lazimi, qui est médecin et militant associatif, je le cite : il faut qu'on soit sûr que tous les moyens de protection seront mises en Oeuvres, or aujourd'hui, même quand l'alerte est donnée par la victime elle-même, il y a des ratés, à à fortiori, on peut imaginer les ratés que pourrait engendrer l'alerte lorsqu'elle ne vient pas de la victime elle-même, c'est pourquoi nous ne pouvons rester au milieu du gué avec cette disposition, il s'agit de l'étoffer pour garantir une aide effective aux victimes de violences conjugales et non les mettre en porte-à-faux, on ne les accompagne, il n'y en pas jusqu'au bout de leur démarche. Madame Cohen Madame la rapporteure pour la vie de la commission si madame. Président donc cet amendement tend à permettent la délivrance d'une ordonnance de protection en cas de levée du secret professionnel ce professionnel aurait porté à la connaissance du procureur de la République, une suspicion de violences conjugales, après avoir levé le secret votre amendement en fait est satisfait par les dispositions de l'article 515 tiré 10 du code civil qui permet déjà au procureur de la République de demandes du Nord de protection avec l'accord de la victime, donc c'est une demande de retrait parce qu'il est satisfait. j'ai une petite incompréhension donc je préfère me poser la question, maintenant c'est le moment, là on est dans le cas du fait que la Perse la victime donc ne souhaitent pas qu'elle est qu'elle est victime de violence etc donc c'est le médecin qui l'informe qu'il va donc passer outre le secret médical, donc on dit on dit oui mais ces satisfait parce que de toute façon l'ordonnance de protection et et déposé à partir du moment où la victime est d'accord, mais là on est dans un désaccord de la victime. Donc on donc ce n'est pas satisfait.

ça va être plus difficile. Il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais donc mettre aux voix l'amendement qui est maintenu par Madame Cohen, avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient l'amendement 80 n'est pas adopté, je mets aux voix, l'article 8 bis. Qui est pour. Qui contre. Qui s'abstient, il est adopté, je mets aux voix, l'article 8. Qui est pour, qui est contre. S'abstient, il est adopté article additionnel après l'article 8 heures un amendement numéro 15 présenté par Madame Benbassa. L'article 8 de la présente proposition de loi prévoit la remise d'un certificat médical constatant les blessures d'une victime de violences, lorsque son examen par un médecin a été requis par un officier de police judiciaire où un magistrat, cet amendement vise à compléter ce dispositif en souhaitant inscrire dans la loi l'obligation pour le médecin qui le reçoit la victime lors d'une première visite de lui remettre un certificat d'examen médical constatant et les blessures qui lui ont été infligés et ce, même lorsque la victime ne s'est pas au préalable présenter aux autorités judiciaires, il semble évident que les victimes de violence, et plus particulièrement celle de brutalité dans un cas d'conjugales sont en droit d'être en possession de leur 1er examen par le personnel soignant d'un document qu'on s'attend la nature et la gravité des coûts qui leur ont été portées notamment dans la perspective de possibles procédures d'indemnisations civiles dans les fêtes, cette pratique est déjà recommandé par la Haute autorité de santé, elle ne trouve cependant pour l'heure aucune consécration législative dans nos textes juridiques, il va donc s'agir par cet amendement de faire concorder la pratique et le droit, comme le préconise, par ailleurs, l'une des mesures issues du Grenelle des violences conjugales, merci. patiente j'ai une patiente arrive et demandent un certificat, un médecin quelle que ce que sa spécialité, même s'il est pas le médecin traitant de la patiente il va rédiger ce certificat en mettant dessus je constate etc et je le remet en main propre pour faire valoir ce que de droit, donc c'est quelque chose qui existe déjà, donc cet amendement en fait est est satisfait. Merci madame la rapporteure monsieur le mini. Merci madame la présidente, ce sera un avis défavorable car si je comprends bien l'intention donc que vous proposez ne peut pas recevoir un avis favorable tout d'abord, rien n'empêche d'une part, à l'heure actuelle, que le professionnel remettent à la victime, le certificat médical initial et c'est d'ailleurs une préconisation de la Haute autorité de la santé après les recommandations de la Haute autorité de santé, de la santé n'ont pas forcément obligé à figurer dans la loi, ça peut être d'ordre réglementaire, mais surtout par ailleurs et surtout la rédaction de votre amendement la fin du texte laisse à penser que le certificat médical préciserait que l'état de santé, le résultat de cette violence ainsi qu'il est rédigé, or vous le savez probablement, madame la sénatrice la déontologie médicale précise. Que le médecin n'a pas à se prononcer sur les dires du patient, les Liens de causalités ou encore la responsabilité d'un tiers déontologie médicale interdit. Aux médecins de faire ainsi, c'est à l'enquête aux enquêteurs à la justice, l'enquête de décider quels sont ses Liens de causalité, non pas au médecin qui lui se borne parce que. C'est son métier, a constaté à décrire les faits suite à un examen de de la victime, voilà donc pour ces 2 raisons, madame, président, ce sera un avis défavorable. Merci monsieur le ministre je et s'il n'y a pas de demande d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement numéro 15, qu'il y a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

monsieur le président. Oui, madame la présidente, c'est un amendement de cohérence rédactionnelle, il est, il est défendu, il modifie l'intitulé du chapitre 7 de la PPL afin de mieux prendre en compte le chien de dispositions qui est qu'il comporte à l'article 9 bis. Merci, cher collègue Madame la rapporteure. Ce complément est utile, nous sommes favorables. Avis favorable Monsieur le bas, excusez-moi, madame la ministre à vie du gouvernement. Pour les mêmes raisons, c'est un avis favorable cet ajout, nous sommes tout à fait justifiée. Merci madame la ministre, je vais donc mettre aux voix l'amendement 75 qui a reçu un avis favorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Ces contres. Qui s'abstient l'amendement 75 est adopté, je mets donc aux voix le chapitre. Ah bon, il est adopté, comme ça, article 9. Nous avons d'abord une prise de parole de Madame Annick Billon. Merci madame la présidente, les articles 9 et 9 bis de la proposition de loi concerne la saisie des armes détenues par une personne suspecte dans le cadre d'une perquisition, cette disposition reflète le constat établi par le rapport de l'Inspection générale de la justice sur les homicides conjugaux, publié en octobre 2019 68 % des agressions ont été commises avec une arme, qu'il s'agisse d'une arme à feu ou d'une arme blanche et pour cette dernière, dans la grande majorité d'un couteau toute évolution de la loi susceptible d'empêcher des agresseurs de détenir une arme et donc une avancée, vous l'avez d'ailleurs signalé madame la ministre, dans votre intervention lors de la discussion générale toutefois la proposition de loi pose 2 problèmes : d'une part, l'article 56 du code de procédure pénale, qui modifie l'article 9 concerne les personnes suspectées de crimes, or le plus souvent les féminicides surviennent après une longue suite de violences psychologiques et physiques qui ne relèvent pas nécessairement d'agissements criminels la menue mesures prévues par l'article 9 n'intervient-t-elle donc pas trop tard dans le parcours de l'auteur de violences, cette disposition est-elle vraiment abouti, ne faudra-t-il pas poursuive ce débat avec le texte suivant : ce ne sera jamais que le 4ème depuis la loi de 2018, d'autre part, comme le rappelle la récente enquête publiée par le journal Le Monde intitulé féminicides mécanique d'un Crime, on compte un certain nombre de féminicides par strangulation ou par défenestration par ailleurs le catalogue des armes par destination auxquels ont recours les criminels et les assassins et sans limite de nombreux hommes ont tué leur femme avec des objets du quotidien, ces remarques me conduisent donc à souligner une nouvelle fois que le texte que que nous d'elle dont nous débattons n'est pas l'Alpha et l'oméga de la lutte contre les violences conjugales, si je me réfère à nouveau récent rapport de l'Inspection générale de la justice, les solutions relèvent aussi et surtout de la généralisation de projets de juridiction ambitieux d'un suivi sans concession des auteurs de violence, de leur éviction systématique du logement d'un contrôle strict des interdictions de contact avec la victime d'une meilleure articulation entre les services de police, gendarmerie et et les parquets et d'un décloisonnement entre les différents services d'une même juridiction les solutions relèvent d'un attirail préventif plus que de la confiscation des armes ces articles représente une avancée importante, mais pas suffisante pour lutter contre la violence, je vous remercie. Merci, cher collègue, je mets aux voix, l'article 9 qui est court. Qui contre. Qui s'abstient, il est adopté au 9 bis, un amendement 81, il est présenté par Madame Cohen. Merci madame la présidente, c'est un amendement de suppression ne vous étonnera pas tant notre pro, notre position sur le sujet, je crois, est tout à fait cohérente au fil de nos débats, lutter contre les violences faites aux femmes, et plus encore vouloir protéger ses victimes ne peut se résumer, je l'ai dit à plusieurs reprises à une surenchère répressive, certes modifié notre code pénal en alourdissant les peines est à mettre en heures, puisque cela a finalement somme toute n'engage aucun moyen supplémentaire, mais on le sait, cela ne va pas dissuader les hommes violents qui ne cesseront sûrement pas de l'être, même si ils encourent une peine éventuellement doubler voire tripler, malgré l'échec le flagrant d'une telle politique menée déjà depuis quand même de nombreuses années, nous ne comprenons pas pourquoi vous continuez notamment chers collègues de droite, comme les membres d'les membres d'ailleurs du gouvernement de continuer dans cette voie, alors que l'article 9 représentent une véritable avancée en permettant aux OPJ la saisie d'armes détenues par les personnes suspectées de violence cet article 9 bis propose de me permettre aux juridictions de prononcer des interdictions relatives aux armes et au contact avec les victimes, en plus d'une peine d'emprisonnement et non pas seulement à la place d'une peine d'emprisonnement dans un contexte, on le sait, de surpopulation carcérale et alors que la majorité de nos voisins européens et surtout ce qui note une récession de la délinquance et des violences en général sont engagés sur la voie de la décroissance carcéral, nous proposons de supprimer des oui pardon, des peines alternatives à l'emprisonnement par cet article, ce qui paraît quand même assez aberrant, je le répète inlassablement pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes, nous sommes convaincus qu'il s'agit de conduire une politique d'éducation et de prévention des violences sur le long terme et je crois que c'est partagé par bon nombre de mes collègues et non d'assembler des dispositions pénales répressive en répétant finalement des erreurs qui ont déjà été commises par le passé, donc nous voulons au contraire nous penser que les meilleures réponses à apporter à cette problématique son nature préventive et en particulier éducative et qu'elles sont à mettre en oeuvre le plus jeune âge en ce sens d'ailleurs, il serait intéressant de faire un bilan, par exemple des dispositifs existants et de ce expérimentés tels que l'ABCD, de l'égalité on préconiser de nouveaux outils pour améliorer les politiques publiques menées en ce sens, donc voilà pourquoi nous faisons cet amendement. Le M. Cohen madame la rapporteure, avis de la commission. Merci madame la la présidente donc ma chère collègue cet amendement entend donc supprimer la possibilité de prononcer des peines complémentaires à l'emprisonnement, nos collègues puis donc la nécessité d'une politique d'éducation et de prévention en matière de violence, donc je suis d'accord avec cette nécessité d'une politique éducative et préventive, bien évidemment, mais en fait, l'article 9 là, cette fois, c'est une vraie avancée dans la protection des femmes il ne supprime pas la possibilité de prononcer des peines alternatives, il les maintient, il prévoit simplement qu'en matière de saisies d'armes datée du de paraître et d'interdiction d'entrer en contact avec la vie. La peine pourrait être pourra aussi être prononcer cumulativement avec une peine de prison c'est cumulatif. Et c'est. Sur ces sujets ponctuels il y apparaît en effet important de pouvoir protéger des victimes pendant et après la détention, donc il ne s'agit pas d'augmenter la population carcérale de mieux protéger les victimes, donc c'est pour ça que je vous demanderai de le retirer, sinon ce serait un avis défavorable. Madame le rapporteur, madame la ministre à vie du gouvernement. Merci madame la présidente, madame la rapporteure, madame la sénatrice pour ce qui nous concerne. L'article 9 bis présente un intérêt majeur pour la protection des victimes, parce que le tribunal pourra en plus d'une condamnation à l'emprisonnement désormais faire interdiction à un conjoint violent de rencontrer la victime pendant une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans, sans pour autant avoir à assortir la peine d'emprisonnement d'un suivi judiciaire comme le sursis probatoire et donc ça se révélera particulièrement utile pour les condamnés absents, notamment à leur compte desquels le tribunal prononce en général peu de mesures de suivi une mesure de suivi étant nécessaire au prononcé de l'interdiction de contact par ailleurs la peine d'interdiction de contact autonomes demeure en peines alternatives à l'emprisonnement, par ailleurs, l'article ne vient donc pas supprimer une peine alternative à l'emprisonnement mais permet qu'elle soit prononcée par le juge non plus simplement en alternative, mais aussi en peine complémentaire et, bien évidemment, tout cela n'empêche pas la mise en oeuvre de politique éducative, même si je partage votre préoccupation sur la nécessité d'en présenter des bilans et le ministre de l'Éducation nationale s'était engagée juste avant le confinement à présenter très rapidement un bilan d'un audit qui l'a mené sur toute l'année écoulée sur les 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle qui sont mises en oeuvre par an depuis l'année dernière, cela a été bloqué par la période de confinement, mais sans nul doute dans les mois qui viendront nous pourrons voir avec le ministre de l'Éducation nationale pour que cet audit soit présenté, et c'est donc un avis défavorable. Merci madame la ministre, madame Cohen. à la lumière des explications que vient de me fournir madame la Mini je vais retirer mon amendement est d'autant que j'ai senti aussi qu'elle était en tout cas aussi préoccupés que que nous sur le côté évaluations bilan donc je pense qu'on aura son soutien, donc ça. Très bien, merci Madame Cohen, l'amendement 80 et retiré je mets aux voix, l'article 9 bis qui est pour. Qui compte. Qui s'abstient, il est adopté, article 10. Madame Billon pour une prise de parole. Merci madame la présidente, cet article tire les conséquences d'un constat désormais classique sur la stratégie de l'auteur de violences, l'utilisation des nouvelles technologies technologie pour enfermer ses proies dans une camisole de force numérique, le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur les violences faites aux femmes en ligne publié en 2018 est très éclairant sur ce danger qui menace les femmes comme les enfants dans les foyers, violents dans le contexte de séparation très conflictuelle, la délégation aux droits des femmes avaient travaillé sur cette dimension des violences dans son rapport d'information intitulé prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société, publié en 2018 le cyber contrôle dans le couple et de hélas classique, un logiciel espion permet au conjoint violent de savoir à tout moment où se trouve sa victime et de tout connaître de sa vie, ça a été tout à l'heure, cité par une collègue de la délégation dans le contexte de la séparation, seul office logiciel installé sur le téléphone portable d'un enfant permet à l'auteur de violences, d'exercer son emprise à distance, sur la mer, donc notre délégation se rouge réjouit bien évidemment que ce texte prenne la mesure d'une dérive qui accroît la menace exercée sur les victimes par des conjoints et des pères violents, je vous remercie. Madame la présidente, nous passons à l'examen de l'amendement 51, il est présenté par Madame de La Gontrie. 51. Je voulais essayer de faire gagner du temps à l'ensemble de nos collègues, puisque le 51 52 53 54 procède du même raisonnement qui est d'étendre aux anciens conjoints on sien concubins anciens partenaires liés par un Pacs. La circonstance aggravante qui est prévu dans le cas de d'une série d'atteinte à la vie privée qui sont à la fois la géolocalisation la violation du secret des correspondances, l'usurpation d'identité et l'envoi de messages malveillants, ce sont donc l'ensemble de comportement, ça a été rapidement évoqué à l'instant par Annick Billon qui peuvent être mises en oeuvre par un conjoint à l'égard. De l'autre et qui sont effectivement très difficile à supporter, sauf que ne sont pas prévues, les anciens conjoints partenaires etc, or nous savons que c'est d'ailleurs essentiellement plutôt après la séparation, que se passe ce type de comportement, alors je pense que l'on me répondra que cette circonstance est déjà prévue par le code pénal n'ont pas les circonstances précises que nous évoquons, mais le fait que, une sanction pénale encourue pour une infraction causée par un conjoint la circonstance aggravante du fait que ce soit posée par un conjoint peut être étendu à l'ancien conjoint, sauf que je pense qu'il est nécessaire dans cet article que l'infraction précise bien vise bien sa cible, à savoir les anciens parce que, encore une fois, ce n'est pas pendant le mariage pendant le Pacs pendant le concubinage que les problèmes les plus violents se passe c'est souvent après et c'est pour cela qu'il faut l'introduire dans cet article. Si cher collègue alors l'avis de la commission sur l'amendement 51. Merci madame la présidente, donc sur le fond, nous ne sommes pas défavorable à cet amendement qui vise à ce que la circonstance aggravante s'applique aussi aux anciens conjoints, concubins, partenaire de Pacs, cependant, comme nous l'avons dit ce matin en commission des lois, il est déjà satisfait par la rédaction de l'article 132 tirer 80 du code pénal, dit loi des ex-des anciens cet article dispose que dans les cas prévus par la loi, le règlement, les peines encourues pour un Crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacs, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas cette circonstance aggravante est également constitué Kant, les faits sont commis par les ex-donc c'est une demande de retrait sinon avis défavorable. Merci madame la rapporteure, Madame la Ministre à vie du gouvernement. Merci madame la présidente, madame la rapporteure, madame la sénatrice exactement pour les mêmes motifs, et comme vous l'avez dit, vous-même madame la sénatrice, nous considérons que c'est déjà satisfait donc, même avec Madame la rapporteure. Merci, s'il n'y a. Pas de demande d'explication de vote je mets aux voix l'amendement 51 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient l'amendement 51 n'est pas adopté, je mais aux voix, l'article 10 qui est court. Qui est contre eux. S'abstient, il est adopté, article 10 bis. Nous avons l'amendement 52 on considère qu'il est défendu madame de La Gontrie, le 52 il est défendu. Oui, d'accord, donc madame la rapporteure, avis de la commission même avis défavorable, madame la même âge mais ma vie, donc l'implant, l'amendement 52 avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, donc il n'est pas adopté, je mets aux voix, l'article 10 bis qui est pour. Qui est contre, s'abstient, il est adopté, article 10 terre amendement 53. Donc défendu même avis de la commission et du Gouvernement défavorable, on est bien d'accord, donc je le mets aux voix le 53 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, je mets aux voix l'article Dister qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, article 10. Waters amendement 54 même de La Gontrie même présentation, même avis de la commission et du Gouvernement défavorable je mets aux voix l'amendement 54 avec l'avis défavorable que la Commission et du gouvernement qui est. Pour qui est contre. S'abstient, il n'est pas adopté, nous passons à l'amendement vingt-trois, présenté par Monsieur Thani Mohamed Soihili. Chers collègues. Merci madame la présidente, Madame Monsieur le Ministre, cet article des squatters. Adopté en commission, introduit dans le code pénal une circonstance aggravante pour les appels téléphoniques ou l'envoi de messages malveillants réitérés parce que la victime et le conjoint, il a sorti ainsi ses faits lorsqu'ils sont commis par le conjoint, le concubin de la victime, ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende

cette infraction est assortie d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ainsi dans une perspective de cohérence et afin de ne pas créer d'asymétrie entre entre ces 2 situations, il est proposé d'aligner par un renvoi les peines pour harcèlement moral entre conjoints et pour appels ou messages réitérés malveillants adressés au conjoint. Collègue madame la rapporteure, avis de la commission. C'est une mesure de mise en cohérence qui est bienvenue, donc c'est un avis favorable. Merci beaucoup, Madame la Ministre vie du gouvernement. C'est madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le sénateur. Pour des raisons purement juridique nous concernant, ce sera une demande de retrait et sinon rejet, je vais vous exposer les raisons du gouvernement l'amendement adopté en commission des lois à créer une circonstance aggravante du délit d'envoi réitéré de messages malveillants lorsque l'auteur est le conjoint ou concubin de la victime portant la peine à 2 ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende, et en l'absence de circonstances aggravantes, ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le texte adopté par votre commission est donc en parfaite cohérence avec l'aggravation par cette proposition de loi de la peine de un à 2 ans d'emprisonnement encouru pour les délits d'usurpation d'identité ou d'utilisation des données personnelles ou encore de la violation des correspondances de la victime par son conjoint, il n'y a pas de raison, selon le gouvernement de vouloir aggraver plus fortement la sanction en reprenant la peine de 3 ans d'emprisonnement prévues par l'article 222 33 Tiret de Tiret un du Code pénal en cas de harcèlement moral au sein du couple nous considérez-vous ces situations sont différentes dans le cas du harcèlement, il doit être démontré que les fermes, je cite, eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale, mais cela n'est pas pas exigé en cas d'appels téléphoniques répétés, il nous semble donc normal que le harcèlement soit plus sévèrement réprimées et s'il est établi que les appels téléphoniques ont provoqué cette dégradation des conditions de vie de la victime, alors dans ce cas, les faits seront poursuivis sous la qualification de harcèlement et pas sous celle de appels téléphoniques malveillants pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, le gouvernement propose le retrait de cet amendement et à défaut son rejet. Merci madame la ministre, monsieur le président, vous avez la parole. Oui, madame la présidente j'ai bien entendu les les motivations de, de, de Madame la Ministre, mais je le précise, il s'agit d'une question de cohérence par rapport à l'échelle des peines, je ne suis pas en train de discuter ce qui peut constituer l'une ou l'autre des infractions, mais une fois le juge

des peines qui va peut-être être réformé, on lui demande à plusieurs reprises, mais en l'état, nous ne voulons pas sortir de cette échelle de peines et ce renvoi

Très bien, chers collègues, nous avons bien compris et donc nous allons mettre aux voix l'amendement 23 qui a reçu un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui compte qui s'abstient l'amendement 23 est adopté, je me voix l'article 10 quater, qui est pour. Qui est contre. S'abstient, il est adopté, article 11.

Parole de du ministre pour un un article important qui porte une disposition importante, comme l'ensemble des dispositions de cette loi, évidemment, mais le Grenelle des violences conjugales, pour la première fois à ce point à appréhender la question des violences conjugales et des violences faites aux enfants de façon conjointe concomitante et c'est effectivement c'était une une nécessité car nous le savons les chiffres nous le démontre, souvent quand il y a violence conjugale, il y a des enfants qui ne sont. Plus témoin qui ne sont pas témoins qui sont de véritables victimes des violences encourus, le sujet de cet article 11 apporte sur la question des faits pédo-criminels. Et je voulais attirer votre attention sur le fait que les victimes de faits de pédocriminalité s'avère être fragilisé tout au long de leur existence et que plus tard dans leur existence dans le rapport aux autres dans le rapport à un conjoint ses victimes vont être. Victime Victime à nouveau à plusieurs reprises, elles vont parfois aussi être auteur et c'est d'ailleurs aussi des grands je pense avancer d'une part du Grenelle et des mesures portées par la secrétaire d'État et les mesures que je porte au sein du plan de lutte contre les violences faites aux enfants de. De s'atteler de s'attaquer également aux auteurs dans une logique de prévention. Avec la mise en place d'un certain nombre de centres de prise en charge des auteurs s'agissant des violences conjugales, telle qu'annoncée il y a quelques 2 jours, je crois, par la secrétaire d'État, et c'est une disposition. également du plan de lutte contre les violences faites aux enfants du 20 novembre dernier que 2 de développer, de mettre en place, pardon, un numéro d'appel. les auteurs potentiels de faits pédocriminels en association avec le Centre de ressources d'intervenir pour les intervenant auprès des auteurs de violences sexuelles, les cris, mesdames et messieurs les sénateurs, la France. Malheureusement, est le 2ème pays européen en nombre de téléchargements de contenus pédo- pornographiques. Chaque année, ce sont plus de 100000 connections téléchargement AD sites. Contenant des images pédo-pornographiques. 100000 auxquels vous pourrez ajouter 50000 supplémentaires qui nous sont envoyés des États-Unis, j'étais hier avec le secrétaire d'État Laurent Nunez pour visiter la plateforme Pharos, chaque mois, ce sont près de 300000 tentatives de connexion sur des sites pédo-criminels bloqués qui ont lieu dans notre pays 300000 chaque mois. Je peux donc vous assurer que la protection des mineurs doit passer par une répression forte des pédocriminels en ligne qui aujourd'hui ont un sentiment d'impunité derrière leur écran s'agit aujourd'hui d'un marché international qui est devenue, pour certaines organisations criminelles, un véritable Business au même type que la drogue ou la contrebande et je rappelle que derrière tout échange d'images. Ou de vidéos Pernod pornographiques. Il y a un mineur agressé, il y a une victime. Il y a dans la pédopornographie inculte de l'inédit. On considère que 20 à 30 % des personnes qui consultent des images pédo-criminels sont aussi des producteurs. D'images. Pédocriminels et que donc, vous avez des enfants victimes derrière ces images, alors la protection de l'enfance en ligne est une condition que sa préservation hors ligne et ce d'autant qu'il existe une imbrication de plus en plus forte, vous le savez, entre activités en ligne et hors ligne aggravé la peine encourue pour les pédocriminels qui consulte habituellement des images pédopornographiques. Les hackers ou les détiennent permettra d'atteindre un objectif auquel je tiens tout particulièrement cela entraînera une inscription automatique au Fijais le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, ce qui n'était aujourd'hui qu'une faculté pour le juge jusqu'à ce jour, l'inscription automatique au Fijais se fait pour les peines encourues de 5 ans de prison la consultation d'images pédopornographiques. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à votre vote ce que votre de la la CMP n'était que de 2 ans et c'était donc au juge de décider. Si l'auteur devait être inscrit au Fijais ce que le juge faisait dans 50 % des cas. C'est-à-dire que dans 50 autres pour 100 des cas, soit à peu près 500 personnes chaque année. Les auteurs de consultation de sites pédocriminels n'était pas inscrit au fichier des agresseurs sexuels et que donc le lendemain, il pouvait être réembauchés auprès d'une structure. Accueillant des jeunes enfants. Par exemple, c'est ce à quoi nous voulons mettre un terme par cet article, cette inscription automatique le sera désormais pour une durée minimum de 20 ans et à l'obligera le condamné a déclaré régulièrement son adresse au commissariat ou à la gendarmerie, cette inscription permettra donc d'éviter que le condamné ne soient recrutés pour exercer une activité en contact avec des mineurs à cet effet, sachez que, par ailleurs, en février dernier avec la garde des Sceaux et la ministre des Sports, nous avons lancé une mission d'audits et d'appui afin de garantir que la consultation du sujet soit systématique par l'ensemble des administrations et par l'ensemble des collectivités locales parce que c'est bien de prévoir des dispositifs, il faut encore faut-il que les administrations les connaissent. Et hier, recours. Voilà, Mesdames et messieurs les sénateurs tout le sens de cet article 11 à auxquels nous tenons particulièrement et je ne doute pas qu'il en est de même pour vous. Monsieur le ministre, je donne maintenant la parole à Madame de La Gontrie, pour présenter l'amendement 55. Merci Merci madame la présidente, le ministre a a parfaitement décrit le mécanisme du Fijais qui est donc ce fichier des auteurs d'infractions sexuelles qui a été créé il y a maintenant quelques années, mais il convient de préciser, c'est l'objet de de l'amendement en tout cas sa motivation qui peut figurer dans ce fichier, la commission a souhaité introduire une inversion du mécanisme puisque il a été décidé, le ministre a a a a fait l'impasse sur cet aspect particulier que lorsqu'il ne s'agit pas de personnes condamnées mais de personnes mises en examen. Elles peuvent nettement en moins être inscrite au Fijais si le juge d'instruction le décide. Et ce qui est proposé par la commission c'est que désormais ce soir le principe se soit l'inscription au Fijais et que le juge d'instruction et simplement la possibilité de ne pas l'inscrire, alors vous allez peut-être trouver que la chose est un petit peu pointilliste mais encore une fois, évidemment le Fijais et très utile, si tant est qu'ils soient consultés. Dès lors qu'il recense les personnes condamnées. Mais là il s'agit de personnes mises en examen. Et donc ça veut dire que pendant les années. Qui vont durer qui vont voir se dérouler les procédures concernées, ces personnes vont rester sur ce fichier et qui y a accès. Les policiers, les magistrats, mais aussi les préfets, les maires, les responsables d'associations, par exemple, peuvent interroger peuvent interroger l'administration pour demander si la personne qu'ils veulent recruter et ou non inscrite au Fijais, donc on voit que le Champ des personnes qui peuvent consulter et extraordinairement vaste. Donc à partir de là, il faut s'interroger sur la pertinence du fichier. On se rassure en indiquant que, bien évidemment, les parquets. Ont l'obligation de retirer les mentions dès lors qu'elle ne serait plus pertinente, nous voilà rassurés, sauf que ça ne se passe pas comme ça, vous avez sûrement souvenir du fichier qui s'appelait le STIC. Dans lequel il y a des millions de Français. La CNIL, quelques années après la création du STIC a constaté que 40 % des informations qui étaient sur ce fichier étaient inexacts donc si j'attire votre attention et si je souhaite que ce soit le juge d'instruction qui décide de l'inscription et que ce ne soit pas un principe intangible et qu'il ne puisse que par exception le refuser, c'est parce qu'en réalité, nous allons donc accepter que des mises en examen non condamnées figurent dans un fichier qui sera accessible. à beaucoup de catégories de personnes pendant des années, très longues et sur lesquels le parquet en réalité parce qu'ils n'en ont pas le temps ne fera jamais le nettoyage, voilà l'objet de mon amendement. Merci madame la présidente, effectivement le le Fijais c'est un outil précieux de prévention de la récidive, il peut en effet être consultés par différents employeurs : l'éducation nationale, par exemple, pour s'assurer que les personnes embauchées ne sont pas poursuivis ou condamnés pour certaines infractions commises sur un mineur ce fichier contient déjà le nom des personnes qui n'ont pas été condamné définitivement, il est également possible, la juge d'instruction d'inscrire sur le fichier, le nom d'une personne mise en examen et placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence sous surveillance électronique, nous avons souhaité favoriser l'inscription de ces personnes sur le fichier, en fait, en faisant de l'inscription de la règle et de la non-inscription d'exception, c'est vrai que ça peut aboutir à ce que des personnes finalement déclarée innocente soit temporairement inscrite sur le fichier c'est exact, s'il faut choisir entre 2 inconvénients, on a préféré cependant plutôt celui-là, au lieu de prendre le risque d'embaucher pour un poste au contact des mineurs quelqu'un sur qui pèsent de lourds soupçons soupçon qu'il ait commis un Crime sur mineur en fait, c'est le principe oui, je sais bien mais on s'est dit : le principe de précaution doit prévaloir, or le principe de précaution, c'est un principe d'action, donc il est inscrit au Fijais donc il appartient au service du casier judiciaire, qui gère le fief de veiller à sa mise à jour régulière nous ajoutons qu'un individu qui figure peut toujours demander l'effacement des données le concernant, voilà, ben il faut lui dire. Et ce. Merci madame la rapporteure. Monsieur merci madame la la la présidente. Code de procédure pénale prévoit qu'actuellement de formes d'inscription des personnes dans le dans s'il s'agit de personnes condamnées l'inscription dans le Fijais et sauf exception pour les délits peu graves, je le disais peine encourue peine encourue hein non pas prononcer peine encourue inférieure à, à 5 ans et dans quel cas les peines encourues au-delà de 5 ans, il est, il est automatique, cette inscription est automatique, s'il s'agit de personnes mises en examen par le juge d'inscription, l'inscription n'est possible à condition qu'il a été décidé un contrôle judiciaire : une assignation à résidence sous surveillance électronique, le rapporteur le disait que si le juge leur donne expressément, telle est l'état du droit à votre commission des lois a adopté un amendement de votre rapporteur rendant dans cette 2ème hypothèse l'inscription automatique, sauf décision contraire du juge, on inverse donc la logique telle que vous l'avez exposé cet amendement, portée par la sénatrice de répondre, il propose de supprimer cette modification alors comme vous le savez je je reconnais me félicite de l'importance de l'utilité du Fijais, c'était tout le sens de mon propos liminaire pour mieux protéger nos enfants, je vous le disais, là aussi, un travail a été engagée avec la garde des Sceaux, dont je salue l'investissement sur le sujet, un travail interministériel pour que se figeait soit plus systématiquement consultés par l'ensemble des administrations, également que, dans certains cas, qui le justifie, depuis la loi du 20 du 14 avril 2016 la loi Villefontaine, le procureur peut d'ores et déjà informé par écrit l'administration des décisions de mise en examen, rendu contre une personne qu'elles emploient veiller à cette sa mise en oeuvre effective doit être une une priorité mais le dispositif existe déjà pour que les administrations soient au courant de cette mise en en examen pourtant cet amendement de suppression ne me semble pas injustifiée. Et ça sera donc un avis favorable à cet amendement en effet rentre par principe automatique l'inscription dans le Fijais des personnes mises en examen, mais qui sont donc présumée innocente, à ce stade. Et ce, quelle que soit la gravité de l'infraction, nous paraît en effet soulevé d'importantes questions de principes tels que madame la sénatrice les a exposés, il est vrai que les juges d'instruction ordonne peu d'inscriptions dans le Fijais. C'est vrai, moins de 200 chaque année et la garde des Sceaux à travers moi, ici, s'apprête à est prête plutôt que s'apprête enfin les prêtre et Elsa prêtera si vous en êtes d'accord, a adressé au procureur une circulaire leur demandant de requérir plus fréquemment cette inscription au Fijais s'agissant des personnes mises en examen, donc en l'état, ce sera un avis donc qui serait favorable à cet amendement de suppression pour les raisons que nous avons exposé. Merci monsieur le ministre je suis saisi de 2 demandes d'explications de vote, tout d'abord Madame V. rien. Merci madame la présidente, alors quant à moi je ne voterai pas cet amendement : à quoi sert le Fijais principalement à éviter d'embaucher des gens qu'on soupçonnerait alors pas forcément encore condamné puisque cela il est évident qu'on ne peut pas les embaucher, mais éviter de les embaucher pour qu'ils puissent travailler auprès de nos enfants est ce que on imagine lorsque un enseignant est soupçonné qu'on va le laisser dans sa classe, alors qu'il est soupçonné, évidemment, il ne doit pas être. Comment renvoyer de l'éducation nationale n'est pas encore condamné mais très clairement, l'éducation nationale va éviter de le laisser dans sa classe, il va bien, le mettent de côté en le gardant mais en évitant un potentiel risque et c'est à ça que sert le Fijais alors non on le consulte pas si facilement, on interroge l'administration qui nous dit : si on peut ou non embaucher la personne après, on n'a pas les détails de la raison pour laquelle on peut ou non embaucher la personne mais très sincèrement, quand vous êtes maire et que vous avez à embaucher quelqu'un pour pouvoir travailler dans un centre de loisirs dans un club de sport. Peu vous importe finalement qu'qui soient soupçonnés ou condamnés déjà soupçonné, vous n'avez pas forcément envie de le mettre au contact de vos enfants, donc c'est voilà ce à quoi sert le Fijais alors après est-ce que là il y a un vrai risque on interfère on on échange le paradigme mais par contre on n'impose pas aux juges. De l'inscrire le juge peut effectivement décidé que, bon, il faut que justice se fasse mais qu'a priori le risque n'est pas suffisant pour inscrire la personne au Fijais mais dans ces cas-là, il le justifie et il prend la responsabilité de remède cette personne auprès des enfants et, sinon, hé bien dans ces cas-là, on protège et c'est quand même important de protéger voilà. Madame veut rien, la parole est à monsieur Alisa. Oui, madame président merci, on est sur un sujet d'une extrême gravité et finalement on, on, on hésite entre 2 bornes entre le principe de précaution et entre la présomption et entre la présomption d'innocence, donc moi en fait, c'est plutôt une question que j'aurais à poser de questions, monsieur le ministre, vous disiez il y a quelques instants que les magistrats finalement ne procéder qu'à 50 % d'inscription, je crois que c'est le le chiffre que vous avez cités, je pense que c'est après condamnation, ce qui me semble extrêmement différents, au regard du principe de présomption d'innocence et j'ai été maire pendant 22 ans, et j'ai malheureusement été confronté à genre de sujet, ça me parle un petit peu quand même, effectivement, on se doit de protéger les les enfants ben des, des, des responsables, que l'on recrute et qui sont chargés de les encadrer, mais pour autant, ce qui me surprend, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on ne fait pas la différence entre la condamnation et entre l'instruction quand on prend par exemple les sanctions en droit du travail, il y a un régime de sanctions, mais vous avez aussi des mesures que vous pouvez prendre à titre conservatoire et là j'ai pas l'impression qu'on fasse la différence entre les 2 et je trouve que c'est quand même extrêmement grave parce qu'effectivement, c'est très grave de maître des enfants en face de délinquants, mais c'est aussi très graves que de faire inscrire dans un fichier, une personne qui, au final, et peut-être aussi innocente, donc j'avoue que je suis très très très perplexe sur la solution à mettre en place et il me semblerait quand même assez judicieux de laisser cette responsabilité aux magistrats. Merci monsieur Alizart, la parole est à monsieur Beuchere. Merci madame la présidente, madame le ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout à l'heure j'étais intervenu pour appeler l'attention sur le principe de cohérence que j'aime beaucoup le principe de préau cohérence tout à l'heure, je le rappelle, c'était : faut-il laisser la liberté aux juges de juger en appréciant toutes les les considérants ou faut-il prescrire au juge des choses plus sérieuses plus directif, parce qu'il juge être il peut se tromper, car la justice est humaine, nous avons parlé tout à l'heure avec madame le Garde des Sceaux. On a fait tout à l'heure dans les amendements que nous avons passé. Des choses qui relevaient d'une logique des choses qui relevaient de l'autre et là encore. Nous, nous prenons les pieds dans le tapis, madame la madame de La Gontrie, je suis obligé de vous le dire tout à l'heure au titre du principe de précaution. Et je ne l'entends parfaitement parce que j'y souscrivaient vous disiez, il faut protéger, principalement les femmes battues, on va dire ça comme cela, et donc on ne sait pas si la personne aujourd'hui et encore, et des condamnés, et donc au type du principe de précaution, il faut protéger les gens et puis cette fois-ci autour du principe de précaution, il ne faut pas les inscrire sur le fichier ceux qui maltraitent les enfants, alors moi je veux bien, soit c'est la présomption d'innocence qui vaut un jour soit c'est le principe de précaution mais quand ne joue d'un argument et de l'autre, alors on fait passer une idéologie, mais certainement pas une cohérence. Merci Monsieur Beuchere alors il n'y a plus à Monsieur le Ministre, pour répondre effet. Question oui, voilà, je vais essayer d'être rapide pour répondre à un certain nombre de des prises de parole alors d'une part bien distinguer effectivement ce qui relève de la condamnation. Et là, il y a bien, inscription automatique, c'est le début de l'article 11 alors que vous vous apprêtez à à voter puisque nous passons la peine encourue de 2 à 5 ans et donc pour les personnes condamnées pour consultation il y aura une inscription automatique au Fijais et donc l'essence, les 50 % deviendront 100 par contre au stade de l'instruction, effectivement, le principe de présomption d'innocence. Toute sa place évidemment. Principe de présomption d'innocence et la liberté laissée au juge de décider d'inscrire ou pas, à ce stade de l'enquête, une personne au Fijais, étant entendu que si le parquet demande cette inscription. Juge d'instruction est obligé. D'inscrire au Fijais la personne et d'y répondre et de et d'inscrire. Une fois encore la loi Villefontaine prévoit qu'à ce stade de l'instruction, le juge puisse prévenir les administrations concernées de la procédure en cours, et d'ailleurs quand nous avons lancé la mission d'audits et d'appui que j'évoquais tout à l'heure avec la garde des Sceaux, tout début février, on se rend compte que, dans l'exemple que vous deveniez madame la sénatrice, l'éducation nationale, il s'avère. Que dans la pratique. S'est développée une culture commune, que vous avez à l'éducation nationale un référent justice que vous savez au sein des académies. parquets des représentants des référents, Éducation nationale et que, de façon assez naturel des cas personnels de l'Éducation nationale, en contact avec les enfants, dans le cas des écoles fait l'objet. D'une instruction tout de suite. Le juge, prévient l'administration et cette personne-là va être écarté du contact des enfants, c'est dans ce sens-là, dans la pratique, loin de tout, tu automatisation du système, à ce stade de l'enquête, où la présomption d'innocence doit encore avoir toute sa place par construction. Que nous voulons agir au niveau des pratiques. Dans chacune des administrations et par ce biais-là pouvoir avoir un système protecteur voilà donc c'est la raison pour laquelle effectivement. Souvent, nous sommes confrontés à devoir mettre en balance des grands principes de notre droit, et la situation, la solution que nous avons trouvé conjointement avec la sénatrice nous semble être équilibré et protecteur de nos enfants et vous vous doutez bien que c'est bien ça qui Kimi à Nîmes, j'espère que vous n'avez pas le moindre doute à cet égard, Monsieur le président. Merci madame la présidente, moi aussi, je voudrais apporter une réponse à ceux de nos collègues qui se sont exprimés et je voudrais d'abord rappeler à notre collègue Pascal Alizart que le code de procédure pénale, que nous avons modifié dans le texte de la commission prévoit déjà que ce sont des personnes mises en examen qui vont être inscrites sur le fichier, donc la mesure de précaution déjà et la seule chose que nous avons fait c'est que dans le texte du code de procédure pénale, il est écrit que l'inscription sur le fichier pour ces personnes mises en examen se fait sur décision du juge et nous avons juste dit que elle se fait, sauf décision contraire du juge, oui, c'est vraiment un déplacement du curseur mais vous posiez la question tout à l'heure, à juste titre, vous affirmiez d'ailleurs la nécessité de laisser la décision aux magistrats bien je vous réponds : la décision reviendra toujours. Au magistrats, nous y avons veillé et cela vide de toute substance l'objection de principe qu'on pourrait faire au texte de la commission, mais comme toujours, quand on discute, il faut revenir au texte pour s'assurer que les choses sont faites correctement voilà, oui, oui, oui, mais justement c'est pour ça que je voulais y répondre parce que la question était légitime et nous nous la sommes posée aussi, et c'est la raison pour laquelle, nous y avons répondu en laissant la responsabilité aux juges simplement le la réponse de principe, c'est que la personne mise en examen qui a commis pas simplement d'ailleurs des agressions sexuelles, mais parfois des agressions criminelles d'une autre nature ou délictuelle, d'une autre nature, à l'égard des mineurs, hé bien cette personne pendant l'instruction, pourra être inscrite et même devra l'être, sauf décision contraire du juge, il me semble que c'est un bon équilibre et compte tenu du fait que les inscriptions au fichier sont vraiment insuffisantes, ce que tout le monde a accepté dans notre débat, je crois que c'est un élément fort pour faciliter la protection de l'enfance parce que c'est vrai, de rue de longs débats pour mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant, à chaque fois que nous avions à prendre une décision dans le cadre de l'élaboration de ce texte de loi, hé bien là aussi on fait passer quand même malgré notre souci de protéger des adultes injustement poursuivi, on fait passer quand même l'intérêt de l'enfant, avant tout, dans le doute, étant entendu qu'il faudra effacer immédiatement du fichier toute personne pour laquelle l'instruction se terminera pour un non-lieu, que ce ne soit pas une tâche qu'on transportera pendant des mois ou des années injustement, voilà ce que je voulais vous dire pour vous apporter une précision, disons donc le si la commission est défavorable à l'amendement de nos collègues, c'est pas parce qu'elle veut faire et la révolution, elle n'en a pas l'habitude, elle ne sait pas encore exercer à ce type de réponse aux problèmes qui lui sont soumis, je vous remercie. je vais maintenant mettre aux voix l'amendement 55 qui a reçu un avis défavorable de quel. La commission est favorable du gouvernement qui est pour.

qui est contre. Qui s'abstient, l'article 11 à est adopté article 11. Une demande de parole de Madame Annick Billon chers collègues. Merci madame la présidente depuis 2014 la délégation aux droits des femmes tentent d'alerter contre l'Exposition croissante des mineurs aux images pornographiques désormais très courante dès le collège, au point qu'on en parle de Génération YouPorn, or la pornographie véhicule une image dégradante des femmes et ne que que que perturber les enfants et les adolescents et entraver la construction de leur propre représentation les codes de la pornographie déshumanise la sexualité en banalisant voire encourageant des relations sexuelles, souvent violentes et mettent à mal la notion de consentement du partenaire de plus, certains spécialistes assimile le traumatisme lié à ces images à celui que cause l'Exposition à des violences donc satisfaction que cette proposition de loi se soit emparé de ce problème, car on ne peut laisser la pornographie faire l'éducation sexuelle de nos enfants, mais la responsabilité des sites pornographiques, bien que nécessaire, ne saurait être suffisante à ce titre, je tiens à rappeler que le rapport de la mission d'information au Sénat sur la prévention, la détection, la répression des infractions sexuelles commises sur des mineurs, plaidait dans sa proposition 11 pour une éducation à la sexualité dans les établissements scolaires, avec une sensibilisation spécifique aux violences sexuelles avec pour présidente Catherine Deroche et comme comme rapporteure Marie Mercier Michel Mosnier et Dominique, rien qui sont dans cet hémicycle, ce soir, ce n'est qu'en alliant le volet préventif au le volet répressif que nous parviendrons à faire évoluer les mentalités chez les plus jeunes et à développer une politique publique efficace et pérenne aussi l'expertise des associations agréées en matière de sensibilisation des enfants et des adolescents au problème des violences sexuelles, est une ressource sur laquelle il est judicieux de s'appuyer cela rejoint notamment une des propositions de cette mission d'information, je vous remercie. Merci, cher collègue, nous passons à la présentation de l'amendement numéro 16 par Madame Benbassa. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État et mes chers collègues. Le présent article 11 un lien entre la consommation de pornographie et les violences qui sont perpétrés dans son cadre conjugal, cette corrélation est pour le moins discutable et hasardeuse, elle s'empare ailleurs fondé sur une. Perception moraliste et puis de la production pornographique, celle-ci n'est pourtant pas toujours uniforme et toutes les productions en la matière ne saurait être perçue comme violente au forcément dégradante pour ses protagonistes féminins et masculins de nouvelles plateformes progressiste amateurs et féministe émerge actuellement dans ce domaine, qui sont loin des stéréotypes oppressif avilissant pour la condition féminine, par ailleurs, nous tenons à rappeler que la 5 prohibition la pornographie ne saurait remplacer des cours d'éducation sexuelle bien architecturé qui seraient dispensés aux adolescents afin que ceux-ci puissent avoir une vision saine et équilibrée de la sexualité, le lien Direct entre la pornographie et les violences conjugales intra-n'étant pas établie et n'ayant d'ailleurs jamais été prouvées, nous estimons que cet article n'a pas sa place dans cette proposition de loi en conséquence c'est en demain en demande la suppression, je vous remercie. Merci madame la présidente, donc, cet amendement vise à supprimer l'article 11 qui a pour objet de codifier une jurisprudence de la Cour de cassation au motif qu'il n'y a pas de lien évident entre accès à la pornographie et les violences conjugales, c'est tout à fait évident, je ne vais pas développer, vous comprenez bien ce que je veux dire, en réalité, la proposition de loi contient, je l'ai indiqué d'un discussion générale des dispositions qui déborde le Champ des violences conjugales et qui s'applique à la protection des mineurs, donc en l'occurrence cet article 11 s'inscrit parmi les dispositions qui visent à protéger les mineurs. Merci, monsieur le Ministre. il est bien question de l'accès par des enfants à des contenus pornographiques, l'article a pour objet de renforcer la législation pour éviter que par un simple clic sur un bandeau où certifie que nous sommes majeurs, un enfant de 10 ans puissent avoir accès à des sites pornographiques, car madame la sénatrice, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui en ligne, les enfants sont constamment confrontés à la sexualité par des contenu sexuel ou pornographique qui le souhaitent ou non l'âge moyen aujourd'hui du premier accès à du matériel pornographique et de 14 ans c'est l'âge moyen très de 50 % des enfants voix du matériel pornographique sur internet pour la première fois à l'âge de 11 ans. Et je suis désolé, l'enfant de 11 ans le cerveau d'un enfant de 11 ans pas fait pour assister à un certain nombre de de ces scènes-là, c'est une forme de violence, moi je le définis comme tels. Les enfants nous disent même qu'ils reproduisent les scènes qu'ils voient. Accédez à pornographie à cet âge-là, ça façonne. Votre conception de la sexualité, ça façonne votre rapport à l'autre, votre rapport au corps votre rapport au consentement et pas que pour les hommes. Pour les femmes aussi. Près de 75 % des enfants nous disent considérer qu'ils ont été exposés pour la première fois du matériel pornographique trop tôt, trop précocement. Par rapport à ce à quoi il pouvait ce Contrairement à, à ce que certains affirment, le sujet des violences sexuelles au sein du couple et la surexposition des jeunes au contenu pornographique, peuvent être considérés comme de sujet tabou, ne sont pas totalement étanches pour les raisons que je viens d'exposer le contact répété précoce des jeunes à ces contenus de toute nature peut avoir des effets sur leur développement, ce n'est pas sans conséquences, je l'ai dit sur leurs rapports sociaux sur leur estime de soi, de la même façon et les rapports entre les les sexes et de nombreux médecins, notamment des pédopsychiatres nous alerte à ce sujet, ça peut modifier leur attitude et leur conception des relations sexuelles et donc, in fine, et être à l'origine de violences sexuelles. Ce renforcement de notre législation doit bien entendu aller de Pair avec d'autres actions que nous mettons en oeuvre, notamment dans le cas du plan de lutte contre les violences que j'évoquais tout à l'heure, le développement de programmes de prévention et d'information auprès des jeunes pour faire émerger chez ces jeunes une pensée critique par rapport à ce qu'ils observent et leur permettent de développer leur propre conception de la sexualité qui puisse se la façonner en temps utile. Seuls par leur propre expérience, mais aussi une meilleure information des parents sur les risques et nous y travaillons avec l'ensemble des acteurs du numérique, notamment suite à la signature d'un protocole de lutte contre l'Exposition des mineurs à la pornographie en janvier dernier avec le secrétaire d'État chargé du numérique Cédric O, ah oui, il y a une demande de parole de Madame Rossignol. Madame Rossignol. Pour dire que je voterai contre l'amendement présenté par Madame Benbassa. Mais que je voulais aussi dire que, pour autant, je ne suis très perplexe sur la l'efficacité de l'article 2 que le gouvernement propose, je ne peux pas lui en tenir rigueur, vous êtes totalement nous sommes totalement désarmés et pour le moment personne ne sait comment empêcher les mineurs d'accéder au matériel pornographique mis à la disposition des adultes, on ne sait pas faire, on peut signé toutes les chartes qu'on veut avec tous ceux qui veulent bien les signer, on ne sait pas aujourd'hui comment faire pour qu'un mineur ne puisse pas accéder à ces sites pour des tas de raisons qui sont liées au fait que ces sites sont très souvent basés à l'étranger et que, et puis que vous l'avez dit, monsieur le ministre avait dû abandonner, je ne veux surtout pas parler de la part de l'accès aux sites pornographiques en général. Mais un jour il faudra bien qu'on se pose la question de savoir ce qu'on pense de cette pornographie qui est aujourd'hui accessible, y compris pour les adultes, bien sûr c'est très toxique pour les enfants, je considère que c'est toxique aussi pour les adultes et que c'est toxique aussi pour les gens qui jouent, je crois que le mot jouer même est est assez indélicat de ma part, les gens qui sont utilisées pour produire ce matériel pornographique. On accepte ça, au prétexte que il s'agit d'affaires entre adultes consentants. Quel consentement des acteurs et actrices de films pornographiques tournés dans à l'étranger dans des pays où il y a aucune régulation ou les gens qui connaissent un peu le sujet dénonce une dégradation constante de la violence des scènes des limites qui sont exposées dans ces films pornographiques qui sont sans limites aujourd'hui, peut-être qu'un jour on pas été dire qu'en fin de compte, la pornographie, fait partie des libertés individuelles. Si Madame Rossignol je vais maintenant mettre aux voix l'amendement 16 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. S'abstient, il n'est pas adopté, je mets aux voix, l'article 11. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient la mort, l'article 11 est adopté. adopté. Article additionnel après l'article 11 amendements 92 rectifié, madame, merci madame la rapporteure au nom de la commission des lois. Merci, merci, madame la présidente, alors c'est un amendement très important, je vais vous présenter maintenant. On a déjà commencé à débattre du sujet que ce soit sur un ordinateur ou sur leur smartphone des mineurs peuvent, de nos jours, très facilement, visionner des contenus pornographiques disponible gratuitement en ligne, ils savent le faire très bien il tape le nom d'un signe. Et ils ont 8 vignettes avec des propositions d'axer tout de suite aux films porno en violation de la loi, de nombreux sites internet ont renoncé à mettre en place un véritable contrôle de l'âge des personnes qui visionne ces images, il suffit d'un clic par lequel le mineur certifie avoir plus de 18 ans, il met juste j'ai plus de 18 ans pour que des milliers de vidéos pornographiques du soit accessible, quelques fois même, on ne propose pas, avez-vous plus 18 ans, quelques fois même, ce n'est pas proposé, pourtant il existe des solutions d'identification de l'âge, par exemple, en passant par France Connect en utilisant une carte de paiement, beaucoup de mineurs visionne ces images dès leur entrée au collège aux intercours, ce qui conduit à s'interroger sur l'impact que la consommation d'images pornographiques pour avoir à moyen terme sur leur développement affectif, psychologique et sexuel, un autre chiffre, on sait que 50 % des moins de 12 ans ont déjà visionné un film pornographique dans sa totalité et que les premières images porno, elles arrivent, je suis pour des enfants de 7 à 8 ans quand il regarde un autre film, tout d'un coup on leur bombardent des images pornographiques à 7, 8 ans, ils ne vont pas forcément s'identifier, donc à la limite, c'est moins grave que à 12 13 ans, bien que ce soit très grave quand même, donc, en principe, l'article 227 Thierry 24 du code pénal permet de sanctionner les sites qui diffusent des images pornographiques susceptibles d'être vu par un mineur la loi existe la peine encourue est de 3 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende mais en pratique, cet article n'est pas appliquée dans l'univers numérique, la justice, elle ne parvient pas à atteindre les éditeurs de ces sites qui sont souvent basées dans des paradis fiscaux très loin et il ne coopère pas avec la France est-ce une raison est-ce une raison la pornographie, c'est un univers particulier la pornographie pour les mineurs, c'est un univers encore plus particulier, les jeunes filles s'identifie aussi avant, c'était plutôt les jeunes garçons, maintenant les jeunes filles aussi s'identifie, on sait que pendant la période de confinement, il y a eu des demandes de de films pornographiques qui ont explosé et encore plus de films pornographiques, violents, comment je vous expliquerai ça simplement autrefois autrefois Xavier les films pornographiques et vous aviez des films pornographiques, violents, c'était une catégorie pour des gens qui étaient sadomasochiste, alors maintenant, dit DDSM enfin, je ne suis pas familière : excusez-moi, avec ça, mais c'était leur droit le plus strict, d'être attirés par des sites pornographiques, violents, on ne partage pas, on essaye de comprendre, sauf que maintenant, avant c'était codifié violent maintenant le violon est devenue dans la pour tous nos graphie, j'ai envie de dire, excusez-moi des de base, ça devient normal qu'une femme se fasse strangulation écartelé et que sais-je, etc mais oui c'est tragique et les petites filles qui vont qui vont voir ça, les jeunes filles qui vont voir ça, elles vont vouloir faire pareil, c'est-à-dire finalement c'est normal le le jeune homme soit violent avec moi : ben non, c'est pas normal du tout, surtout quand on est en construction comme comme cela a été expliqué tout à l'heure donc, cet amendement que je vous propose, avec vraiment j'ai envie de dire, passion et enthousiasme, il propose d'instituer une nouvelle procédure destinée à obliger les éditeurs de ces sites pornographiques à mettre en place un contrôle de l'âge de leurs clients, d'abord, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel leur adresserait une injonction de se mettre en conformité avec la loi, la loi existe, puis il pourrait saisir le président du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il ordonne aux opérateurs de rendre impossible l'accès à ces sites, qui ne pourrait donc plus être consultés depuis la France, on vous propose enfin une action même si on sait que ce n'est pas aussi facile que ça, mais au moins, c'est le début du commencement de quelque chose, ce dispositif, il s'inspire de celui qui est mis en place pour lutter contre les cercles de jeux en ligne illégaux qui repose sur le contrôle exercé par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, ça marche pour les jeux en ligne : pourquoi ça marcherait pas sur les sites porno l'adoption de cet amendement permettrait de mettre en oeuvre et l'engagement que le président de la République avait pris le 20 novembre 2019 lors d'un discours prononcé à l'UNESCO, le président de la République avait donné 6 mois aux acteurs de l'internet pour mettre en place un contrôle parental par défaut, sans quoi il serait nécessaire de légiférer ont les 6 mois, ils sont passés ces faits, les 6 mois on a là une accroche dans la loi pour répondre à l'exigence du président de la République, c'est quand même bien cette question devrait être traitée dans le cadre de l'examen du projet de loi de réforme de l'audiovisuel mais qui est remis aux calendes grecques, on sait très bien que ça ne va pas avoir lieu dans les mois qui arrivent cet avenir, il y a certains, ça va être au mieux en 2021, donc ça ça incite à aborder à l'occasion de cette proposition de loi ces dispositions qui vont véritablement protéger les mineurs, vous allez me dire, les sites qui sont à l'étranger, on va enfermer, il va sans se nourrir de dans la foulée. Peut-être, mais c'est pas une raison pour ne pas le faire, c'est là, vous savez c'est la la fable du petit colibri, il y a un tout petit bec il y a une goutte d'eau pour éteindre l'incendie, dans la jungle, mais il fait sa part il porte sa part : nous avons la responsabilité de faire quelque chose, on ne peut pas accepter de dire on ne peut rien faire quand j'ai été élu maire en 2001, je suis allé à la Maison des ados, on m'a dit : Madame le maire il un souci, il y a des ordinateurs, regardez nos jeunes où ils vont, comment on va faire 2001, c'était il y a 19 ans, là j'ai expliqué aux jeunes à l'époque, il avait 13 ans, qu'il fallait pas qu'ils aillent là-dessus très désigne 13 et 19 32, ils sont 32 ans maintenant ces jeunes-là et ils ont le même problème avec leurs enfants, on n'a rien fait l'univers numérique de nos enfants nous dépasse, on ne peut pas accepter d'être dépassé, on a la possibilité d'avoir une accroche ici je crois vraiment qu'il faut qu'on la saisisse tous ensemble pour protéger nos enfants. Merci madame la rapporteure alors Monsieur le Ministre. Avis du Gouvernement. C'est le gouvernement va essayer d'être aussi. Passionné. Pénétrer que Madame la la rapporteure. Vous, ben écoutez laisse. à vos propres interprétations, vous avez raison Madame Rossignol je vais vous répond Madame la rapporteure, vous avez raison, la seule dispositions de l'article 11 ne suffit pas. à lutter contre ce fléau qu'est l'accès des mineurs à la pornographie, mais c'est un ensemble de mesures. Que nous mettons en place. Pour que chacun des leviers en ciblant parfois les hébergeurs. Parfois, les fournisseurs d'accès, parfois, les éditeurs de contenus, les plateformes, les réseaux sociaux pour qu'à chaque niveau, nous essayons de restreindre d'interdire l'accès des mineurs à la pornographie et Madame la rapporteure, vous avez raison de citer le président de la République et le discours qu'il a effectuée devant l'UNESCO, à l'occasion du 30ème anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant, à l'occasion de la présentation du plan de lutte contre les violences, car la question de l'expédition des mineurs à la pornographie est un sujet qui préoccupe très fortement le président de la République, alors première outil vous l'avez évoqué je l'ai évoqué tout à l'heure, ce protocole d'engagement qui a été signé en présence de Cédric O, secrétaire d'État au numérique avec l'ensemble des acteurs, c'est la première fois que nous mettons autour de la table l'ensemble des acteurs, des associations, évidemment, les fournisseurs d'accès. Les grandes plateformes. Mais aussi les constructeurs de téléphones, bref l'ensemble de la chaîne de valeur car nous pensons que c'est de la responsabilité de chacun. De pouvoir restreindre cet accès des mineurs à la pornographie. Effectivement, vous l'avez rappelé en janvier dernier, ils se sont engagés sous 6 mois la crise était passé par là pour être très honnête, les travaux continués nous avons pris un peu de retard et nous nous sommes donnés rendez-vous au début de l'été. Sous 6 mois pour être en mesure de nous proposer un dispositif, nous leur avons laissé la liberté des moyens, nous avons fixé un objectif : restreindre très fortement l'accès des mineurs à la pornographie, donnez-nous proposez-nous les moyens d'y arriver avec effectivement le contrôle parental par défaut qui nous semblait être, mais ça reste ouvert. Un moyen d'action efficace pour restreindre cet accès si je peux me permettre Madame la rapporteure le l'adoption de cet amendement ne mettra pas un terme et ne mettra pas ah bah cet engagement, la part de l'ensemble des acteurs cet engagement reste nécessaire et nous continuons à suivre leurs travaux qui sont menés sous l'égide du CSA et de l'Arcep 2ème dispositif brièvement l'article 1 de la loi Avia. Que vous avez adoptées et qui a intégré la question de l'Exposition à la pornographie des mineurs, comme un des champs de compétence de cette loi 3ème élément cet article 11 que vous vous apprêtez à voter qui donc réintroduit dans le droit dur une jurisprudence de la Cour de cassation, vous l'avez évoqué qui dit que les simples Disclaimer ne suffisent pas. Comme garantie à ce que les mineurs puissent accéder à un site, et puis l'ajout de Madame la rapporteure, qui confie au CSA la possibilité effectivement de saisir de saisir le juge étant entendu que le projet de loi audiovisuelle, vous aurez l'occasion peut-être de débat, peut-être sous une forme un peu différente, je ne sais pas, je ne veux pas préjuger de l'avenir de ce qui était prévu initialement, mais prévoyez vous le savez, la fusion du CSA et de de l'Arcep, avec la création d'une nouvelle instance, l'art, comme nous, nous avions prévu et nous prévoyons toujours que la question de la lutte l'accès à la pornographie pour les mineurs, fasse partie des champs de compétence voilà donc c'est un ensemble de dispositifs auxquels l'amendement de la rapporteure apporte sa Pierre, fort utile qui je l'espère Madame Rossignol permettra de restreindre très fortement l'accès des mineurs à la pornographie nous faisons pour laquelle la vie sera favorable. Si Monsieur le ministre, s'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement qui a été présentée par Madame le rapporteur avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour. Des contres. S'abstient l'amendement 92 rectifié est adopté, nous passons à l'examen de l'amendement 17 rectifié, il est présenté par Madame Benbassa. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, selon une étude menée il y a 2 ans par le ministère de la Santé et des solidarités, il estimait que chaque année. 170000 enfants sont témoins de violences conjugales intrafamiliales perpétrées dans les foyers français pour le Femina les conséquences néfastes d'une telle Exposition sur le long terme ne sont plus à démontrer, des femmes Drôme de stress post-traumatique et des effets préjudiciables à leur développement cognitif et émotionnel, sont notamment à déplorer, certains en viennent même malheureusement à perpétuer ces schémas comportementaux violent, une fois l'âge adulte atteint, il semble donc nécessaire de reconnaître les traumatismes et les souffrances endurées par ces enfants actuellement sur le plan pénal en moins qu'il n'ait lui-même directement, fait l'objet de violences, l'enfant ne peut être considéré comme une victime à part entière des brutalités intrafamiliales pourtant l'Exposition du mineur aux violences conjugales relève indéniablement de mauvais traitements qui lui auraient été infligées, il est donc nécessaire que le droit pénal français admettent que le préjudice moral et physique qui touche le parent violenter se répercute également sur l'enfant, qui assistent à ces scènes ainsi est-il proposé dans le présent amendement de reconnaître, par extension, que les mineurs exposés aux violences conjugales sont également des victimes directes de ces maltraitances, je vous remercie. Bah, ça, la parole est à madame la rapporteure pour l'avis de la commission. je partage bien sûr l'idée générale qui sous-entend cet amendement, le mineur exposés aux violences en est indirectement la victime, il peut en éprouver un traumatisme qui va le marquer durablement, il peut aussi parfois reproduire une fois adulte, la violence à laquelle il a assisté parce que c'est ce qui connaît j'observe cependant que le code pénal prend déjà en compte cette dimension, les faits de violence au sein du groupe sont en effet punis plus sévèrement quand un mineur a assisté aux faits, donc l'adoption de cet amendement n'entraînerait aucun alourdissement de la peine encourue, donc on peut considérer que cet amendement est satisfait en fait. Si Madame le rapporteur monsieur le ministre à vie du gouvernement. Merci, merci, madame la la présidente, juste avant de donner l'avis du gouvernement et les raisons pour laquelle mon avis sera défavorable juste préciser que ces ces projets de loi audiovisuelle prévoyait le rapprochement de l'Hadopi et du CSA, et non pas de l'Arcep et du CSA, je ne voulais pas oui c'est une annonce un scoop qui n'avait pas lieu d'être voilà petite précision qui a été fait, une fois ceci fait reconnaître évidemment qu'un et un enfant exposé des violences conjugales peut-être traumatisé par celle-ci, être considérés comme des victimes de ces faits, à côté de la personne, le plus souvent sa mère qui, elle, a aussi été victime directe pour autant Madame la sénatrice, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre et violences sexuelles et sexistes a déjà expressément reconnu la qualité de victime de ces mineurs en prévoyant de retenir comme circonstance aggravante des violences conjugales, le fait pour un mineur d'assister à ces violences, l'objectif poursuivi par cette disposition est à la fois d'aggraver la répression est également de permettre de se constituer partie civile du reste dans la circulaire du 9 mai 2019 qui est relative à l'amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes, nous avons donné pour instruction au parquet de systématique, la garde des Sceaux a donné pour instruction au parquet de systématiquement retenir cette circonstance aggravante, je cite, compte tenu de la coloration particulière qu'elle donne au fait et la garde des soins, a indiqué que, je cite encore la d'initiation d'un administrateur ad-hoc devra par ailleurs être envisagée afin de permettre aux mineurs de se voir reconnu comme une victime des faits par ailleurs votre amendement soulève une importante difficulté juridique Madame la la sénatrice en effet n'est constitutionnellement pas possible de créer un délit spécifique d'Exposition des mineurs à des violences conjugales, alors même que depuis la loi du 3 août 2018, ce que j'ai précités, les violences conjugales commises en présence d'un mineur sont aggravées, a même fait ne peut en effet constituer à la fois un délit autonome et la circonstance aggravante d'un autre délit car cela règle cela viole bien connue de non il bis in idem dans le je rappelle enfin que les travaux menés dans le cadre du du Grenelle, contre les violences conjugales, sous la responsabilité de la secrétaire d'État et du plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants sous ma propre responsabilité ont démontré la nécessité de renforcer les unités d'accueil et d'écoute spécialisée pluridisciplinaire pour recueillir la parole du mineur, les yeux à peine et au sein de son plan de lutte contre les violences, présenté en novembre dernier, ses unités d'accueil médico-judiciaire pédiatriques on appelle désormais unité d'accueil pédiatrique pour l'enfance en danger vont être généralisés à l'ensemble du territoire d'ici 2022 madame de la Gondry grâce à l'allocation de moyens supplémentaires, nous avons 64 unités aujourd'hui l'objectif est d'en avoir 104 d'ici 2022, il est prévu que l'audition des mineurs par ces structures à l'issue de laquelle une prise en charge psychologique pour intervenir pourra évidemment concerné les mineurs victimes, témoins, victimes de violences conjugales. Merci monsieur le ministre, je vais donc mettre aux voix l'amendement 17 rectifié, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre.

2 amendements identiques de rétablissement, je commence par le 56 qui est présenté par Madame de La Gontrie. Merci madame la présidente, nous nous préoccupons de savoir comment est-ce que les victimes de violences conjugales, vont pouvoir se faire protéger par la justice et donc engager des procédures notamment l'ordonnance de protection, mais pour cela il faut le plus souvent être assisté d'un professionnel, en l'occurrence d'un avocat, voir, on a évoqué cet après-midi d'un huissier, et donc pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle, à l'Assemblée, des travaux très importants ont été menées conjointement par Naïma Moutchou et Philippe Gosselin qui avait conclu sur l'aide juridictionnelle, et qui avait conclu que dans le cas des violences conjugales, il fallait proposer qu'elle soit attribuée en urgence, sans conditions de ressources dès le dépôt de plainte lorsque le texte dont nous nous occupons aujourd'hui est venue en discussion, il a été prévu, dans un article 12 qui a été supprimée par la commission des lois et que je propose de rétablir que il soit possible d'attribuer lorsque la procédure présente un caractère d'urgence, qu'il soit possible d'attribuer l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, elle devient définitive lorsque le dossier a été instruit pour voir si la personne ne peut réellement bénéficié de la juridictionnelle. La nécessité, évidemment, on le voit bien, c'est-à-dire qu'une personne puisse d'emblée être assisté, curieusement, la commission des lois a décidé de supprimer cette possibilité en arguant du fait qu'il était toujours possible d'obtenir de l'aide juridictionnelle en urgence, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour avoir l'aide juridictionnelle, il se déroule entre 15 jours et 6 mois selon les bureaux d'aide judiciaire de par la France, parce que c'est chaque tribunal qui attribue l'aide juridictionnelle, il y a 2 donc une incroyable hétérogénéité à la fois de délai mais aussi d'objets car chaque bureau d'aide judiciaire et, plus exactement, les tribunaux, les présidents des tribunaux décident en fonction de leur propre jurisprudence selon que l'urgence est est déclaré ou non, et donc il nous a paru et c'est l'objet de l'amendement, il nous a paru très sain que l'on fixe le cadre dans lequel oui on peut demander l'aide juridictionnelle d'urgence de prévoir que ce soit dans des matières qui soit fixée par décret en Conseil d'État, de manière à ce que sur l'ensemble du territoire français les dispositions soient égalitaires. Et donc ça, nous sommes très important, d'autant que j'ai le souvenir d'un échange avec le président en commission. C'est une erreur de penser qu'on peut avoir l'aide juridictionnelle en 24 heures. Il y a une circulaire de la garde des sceaux qui indique à ses bureaux d'aide judiciaire qu'il faudrait que ce puisse être fait en 24 heures en cas de violence conjugale. Mais ce n'est pas la réalité du tout. Donc, encore une fois. Renforcer l'aide juridictionnelle provisoire, c'est très important dans ces matières, et c'est pour ça que nous demandons le rétablissement de l'Arctique qu'il le prévoyait et qui était issu du texte voté à l'Assemblée nationale. La parole est à Madame Cohen pour défendre l'amendement identique 82. Oui, donc c'est un amendement identique donc une explication plutôt proche et moi je suis assez étonné que il n'y ait pas il y a cette attitude-là de de la commission parce que on sait par pertinemment que les les compagnons qui sont violents ont aussi comme attitude pour un certain nombre d'entre eux 2 d'enfermer leurs victimes en fait dans une grande dépendance économique donc je je ne comprends pas que cet aspect-là des choses ne soient pas pris en compte dans ce cas particulier qui en rajoute encore au niveau donc des violences qui sont infligées aux femmes, et d'ailleurs, le rapport d'information de la délégation droits des femmes de l'Assemblée nationale en janvier dernier, estimé que cela faciliterait le parcours judiciaire des victimes de violences conjugales et leur permettrait d'avoir un accès facilité un avocat précisant également, comme le signale d'ailleurs aussi le magistrat : Édouard Durand dont on a pas mal parlé ce soir que cette aide juridictionnelle provisoire doit être ouverte dès le début d'une procédure, soit au moment du dépôt de plainte soit l'enclenchement d'une procédure civile, une telle évolution permettrait à la victime de bénéficier d'une aide appropriée pour s'engager de la manière la plus efficace possible dans cette procédure, elle serait par exemple l'épauler pour se préparer à une éventuelle confrontation pourrait en outre. être domicilié chez son avocat, le temps de la procédure pour toutes ces raisons, nous proposons dans un 1er temps le rétablissement de l'article 12, telle que le proposait les députés Couillard et Gouffier Cha, je vous remercie. pourquoi, en fait, la Commission a fait le choix de supprimer cet article qui propose d'automatiser l'attribution à titre provisoire de l'aide juridictionnelle mais vient en contrepartie limiter le bénéfice de cette attribution provisoire à certains contentieux énumérées par décret en Conseil d'État, elle a estimé que cet article ne présenter qu'un apport très modeste au regard de la situation existante, étant rappelé que la solution dépend avant tout de l'organisation des bureaux d'aide juridictionnelle image et de la manière dont il traite de manière prioritaire les dossiers des victimes de violences conjugales, la circulaire publiée le 28 janvier 2020 par la garde des Sceaux, appelle ainsi les belges à mettre en place un circuit spécifique permettant l'attribution sous 24 heures de l'aide juridictionnelle au profit de la partie demanderesse dans le cadre des ordonnances de protection, ce faisant, les bâches peuvent accorder directement l'aide juridictionnelle à titre définitif ce qui accorde plus de sécurité aux demandeurs qu'une admission à titre provisoire qui peut ensuite être remise en cause au regard de ses ressources, donc la victime elle aura de toute façon un payer l'avocat, pour simplifier, la commission a préféré s'en tenir au système actuel qui donne suffisamment de souplesse aux juridictions et au barrage pour permettre de traiter toutes sortes de situations dans lesquelles l'admission à titre provisoire est nécessaire, les juridictions, on peut en faire usage, lors de la crise du Covid 19 lorsque certains bah j'était fermé, l'article 12 vise à améliorer l'admission à titre provisoire des femmes victimes de violences conjugales, mais ce faisant, il remet en cause tout le système d'attribution de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire actuel en privant les juridictions judiciaires et administratives de leur faculté de l'attribuer au regard de l'urgence de chaque situation sans avoir à se limiter à telle ou telle type de contentieux, voilà pourquoi l'avis est défavorable. Merci madame la présidente, madame la rapporteure mesdames les sénatrices. En ce qui concerne le gouvernement, pour nous, c'est un avis favorable et je voudrais vous expliquer pourquoi l'article 12 renvoie à un décret, la liste des procédures qui permettent d'octroyer l'aide juridictionnelle provisoire parmi ces procédures, les violences conjugales, figure évidemment en première place, mais il nous paraît préférable de renvoyer au décret pour ajuster plus aisément le périmètre concerné par l'aide juridictionnelle provisoire cette disposition, elle vient compléter en réalité une autre disposition, entrée en vigueur au 1er janvier de cette année, qui concerne les juridictions signataire de conventions avec les barreaux en matière d'aide juridictionnelle ces conventions, elle donne lieu au versement de dotations complémentaires, selon les procédures lorsque le barreau mettent en place une permanence d'avocats, or le périmètre de ces conventions intègre désormais les ordonnances de protection donc la réécriture du régime de l'aide juridictionnelle provisoire complémentaire de cette modification du régime des conventions locales va, selon l'avis du gouvernement dans le bon sens et c'est la raison pour laquelle nous proposons un avis favorable pour. Merci madame

qui est contre Qui s'abstient, il n'est, il ne sont pas adoptés. Après l'article 12 un amendement 57, il est présenté par Madame Rossignol. Comme il s'agit d'une demande de rapport, je vais faire vite mais l'idée dans cet amendement, c'est de proposer au gouvernement d'avoir un jour un débat consacré à l'aide juridictionnelle, vous savez que l'aide juridictionnelle est la condition de l'égalité d'accès à la justice pour tous les citoyens et qu'elle est aujourd'hui soumise à beaucoup de questions, en particulier dans les modes de rémunération différenciée dans les montants dans les plafonds de ressources pris en compte et dans un moment où la juste l'accès à la justice semble souvent difficile à beaucoup de justiciables, il serait utile que le gouvernement Vienne un jour à débattre avec nous de ce non pas de ces projets n'ont pas de ces annonces n'ont pas de ces plans, mais de ce qu'il croit ce qu'il faut faire et ce qu'il veut faire en matière d'aide juridictionnelle. Madame Rossignol, avis de la commission madame la rapporteure. s'était opposé à une réforme adoptée au détour d'un amendement à l'Assemblée nationale, donc ceci étant dit, vous ne serait pas surpris, je vous propose l'application de la jurisprudence habituelle de la commission sur les demandes de rapport, c'est donc un avis défavorable. Merci madame la rapporteure, madame la ministre à vie du gouvernement. Merci madame la présidente, madame la rapporteure, madame la sénatrice. Nous sommes évidemment à votre disposition pour un débat sur l'aide juridictionnelle, mais en ce qui concerne ce rapport d'abord je voudrais préciser qu'un 1er rapport parlementaire a été publié l'été dernier et d'ailleurs, le Conseil national de l'aide juridique a produit en 1er rapport précisément sur ce sujet, l'année dernière et une commission a été mise en place, présidée par Dominique Perben et qui doit prendre des premières propositions sur ce sujet d'ici quelques semaines, et ce sera à cette occasion, probablement le moment d'en débattre et c'est pour toutes ces raisons que le Gouvernement émet un avis défavorable. Qui compte qui s'abstient, il est adopté, après l'article 12 bis, nous avons 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune nous commençons par le 9 rectifié présenté par Monsieur Merci madame la présidente, la loi de juillet 91 relative à l'aide juridique prévoit que les étrangers en situation irrégulière peuvent, je cite, à titre exceptionnel, se voir accorder l'aide juridictionnelle, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt je souligne, parce que c'est une conception quand même assez vague dignes d'intérêt. Les bureaux d'aide juridictionnelle on vient d'en parler, dispose ainsi d'un très large pouvoir d'appréciation et selon le défenseur des droits, les pratiques de ces bureaux présente de telles disparités dans le traitement des demandes que l'effectivité de l'accès au tribunal n'est pas garantie de façon uniforme sur l'ensemble du territoire et cette situation est notamment préjudiciable aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales qui, en raison de leur situation irrégulière disposent de faibles ressources et qui ont besoin particulièrement d'être aidé et assisté pour des problèmes de langue et de connaissance du droit afin d'éviter cette différence de traitement, il est utile de clarifier les règles devant être appliquée par ses bureaux et le présent amendement vise à faire en sorte que la situation vécue par une victime de violences familiales soient systématiquement considérés comme dignes d'intérêt. Merci monsieur. La parole est à Madame Benbassa pour présenter l'amendement 18 rectifié. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, plusieurs associations d'aide aux personnes migrantes notamment la Cimade nous ont alertés sur la double peine que subissent les femmes étrangères sur notre territoire, elles sont régulièrement victimes de violences conjugales sexistes et sexuelles mais, contrairement à celles qui sont de nationalité française, nombre d'entre elles ne peuvent s'adresser à la justice, faute de moyens financiers et d'accès à l'aide juridictionnelle en effet les personnes étrangères ne bénéficient pas automatiquement de l'aide juridictionnelle, qui n'est en principe accorder que sous condition d'être de nationalité française ou d'avoir ses papiers de séjour en règle pourtant l'article 3 de la loi sur l'aide juridique, datée du 3 juillet 1991 a ouvert la voie à un élargissement de son attribution ainsi certaines personnes migrantes en situation irrégulière, notamment celles présentes en centre de rétention administrative peuvent-elle en bénéficier, ce n'est pour l'heure pas le cas des étrangères victimes de violences conjugales de harcèlement moral de viols ou d'agressions sexuelles dans les droits ne sont ouverts qu'en cas de régularisation de leur situation, cette position du droit sans particulier allemands inique puisqu'elle laisse les femmes étrangères, dans une situation de précarité de danger à la merci de leurs agresseurs ainsi est-il proposé par le présent amendement de garantir un accès à l'aide juridictionnelle à toutes les personnes étrangères victimes de violences dans le cas de procédure civile, pénale ou administrative et ce, sans condition de nationalité ou de régularité du je vous remercie. si personne n'y voit d'inconvénient et s'il n'y a donc pas d'observation, il en est ainsi décidé et donc nous passons maintenant à l'avis de la commission madame la rapporteure. donc ces amendements 9 et 18 ans fait sont satisfaits par la rédaction actuelle de l'article 3 de la loi du 10 juillet 91, les étrangers peuvent déjà être admis à l'aide juridictionnelle, sans condition de résidence lorsqu'ils sont partie civile dans un procès pénal ou qui bénéficient d'une ordonnance de protection, il n'y a donc pas besoin d'énumérer de manière précise certaines infractions, donc c'est une demande de retrait puisque ces satisfait. Merci madame la rapporteure, Madame la Ministre à vie du gouvernement. Merci madame la présidente, madame la rapporteure, madame la sénatrice Monsieur le Sénateur. Pour les mêmes raisons, et, et, plus précisément, si l'âge ici est entièrement dépendante économiquement et qu'elle ne disposent pas de ressources, hé bien automatiquement, elle est admise à l'aide juridictionnelle, mais le recours à l'aide provisoire permet de mais en plein de mettre en place par très rapidement une assistance par un avocat, donc la rédaction de l'article proposant la proposition de loi nous paraît par conséquent plus sage et peut-être juridiquement plus solide et donc pour ces raisons, nous émettons un avis défavorable.

donc je mais on voit l'avant l'amendement 9. Ratifier qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté après l'article 13 un amendement 10 rectifié bis de Monsieur Young. Merci madame la présidente, il s'agit toujours du problème de la protection des étrangers en France et cet amendement vise à compléter le dispositif de protection des victimes de violences familiales, de nationalité étrangère, ce dispositif a été renforcé en 2016 et 2018 il s'applique aux conjoints de Français titulaires d'une carte de séjour, les conjoints temporaire portant la mention vie privée familiale, il s'applique également aux conjoints de Français titulaires d'une carte de résident aux bénéficiaires d'une ordonnance de protection, un certain nombre de victimes de nationalité en étrangère en revanche ne sont pas protégés il s'agit des conjoints de ressortissants communautaires des conjoints de réfugiés des conjoints de bénéficiaires de la protection subsidiaire donc le présent amendement vise à remédier à cette situation en prévoyant que ces victimes conservent leur type de séjour bénéficie du renouvellement de leur titre de séjour en cas de rupture de la communauté de vie. Merci, cher collègue Madame la rapporteure, vous avez la parole. Donc que votre amendement, mon cher collègue, vise à accorder au conjoint étranger d'un étranger ayant un droit au séjour spécifique, c'est-à-dire un ressortissant communautaire, un apatride, un réfugié ou un ou un bénéficiaire d'une protection subsidiaire : le droit de voir son titre maintenu en cas de rupture de la vie commune, du fait de violences conjugales en temps normal, l'étranger titulaire d'une carte de séjour doit être en mesure de justifier qui continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte s'ils cessent de remplir l'une de ces conditions alors il risque un retrait en l'espèce, bénéficiant du titre de séjour en tant que conjoint l'étranger doit normalement pouvoir justifier d'une communauté de vie affective effective avec son conjoint, certains dispositifs prévoit expressément des exceptions à cette condition de communauté de vie effectifs en cave, on se conjugale, justement, c'est le cas des cartes de séjour temporaires, vie privée et de cartes de résident conjoints de Français et de carte de séjour temporaire regroupement familial mais en l'espèce, rien n'est prévu, si ce n'est parfois à titre réglementaire pour les conjoints de ressortissants communautaires, c'est l'article R. 121 l'amendement donc de Monsieur Dion, notre collègue est donc bienvenue pour harmoniser le traitement de ces cas, quel que soit le titre accordé et exclure le retrait en cas de cessation de la communauté de vie en cas de violence conjugale, c'était un petit peu compliqué, donc j'ai lu avec attention, c'est donc un avis favorable. Merci madame la rapporteure, Madame la Ministre. Si madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le sénateur. En ce qui concerne le gouvernement, la garde des Sceaux a souhaité préciser que le contenu, c'est un moment était, selon elle, déjà satisfait en l'état actuel du droit, en ce qui concerne les conjoints de citoyens de l'Union européenne et puisqu'il convient de préciser que leur droit au séjour n'est pas assujettie à une condition : une communauté de vie mais au maintien du lien marital et cette absence d'exigibilité d'une communauté de vie a été confirmée par une large jurisprudence communautaire et l'amendement numéro 10 aboutirait assez paradoxalement par une lecture, a contrario, a ajouté une condition de maintien de vie commune qui n'est pas prévu par la directive Dominique 38 CE dans les articles L 121 3 et L 122 en sur la transposition en droit interne, en outre, l'article R-121 cela 8 prévoit que le conjoint du citoyen de l'Union conserve son droit jour malgré la dissolution du lien conjugal, lorsque les situations particulièrement difficile exige et je cite notamment lorsque la communauté de vie a été rompu à l'initiative du membre de famille en raison des violences conjugales que ce membre a suivi donc en ce qui concerne les conjoints des étrangers reconnus réfugiés aucune disposition du Ceseda ne permet de retirer la carte de résident délivrée au conjoint dans une réfugiée au motif que la rupture de sa vie commune avec le dit ou la dite ressortissants le renouvellement du titre en cas de rupture de la communauté de vie pour violences et donc d'ores et déjà garanti en l'état actuel de la législation, le droit au séjour des conjoints et des partenaires de protéger subsidiaire et apatrides, victime de violences conjugales ou familiales et lui protégé par la jurisprudence qui exige que l'on tienne compte des violences qui nous ne s'il a pu faire l'objet de la directive 2011 95 du 13 décembre 2011, s'oppose à la rédaction proposée par l'amendement qui placerait le préfet de fait en situation de compétences liées et donc pour toutes ces raisons, au nom de la garde des sceaux, le gouvernement demande le retrait de cet amendement et, à défaut, y sera défavorable. Merci madame la ministre, si il n'y a pas de demande de prise de parole, je mets aux voix l'amendement 10 rectifié bis qui a reçu un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour.

Merci madame la présidence, c'est toujours dans la même dans la même veine de le problème des étrangers victimes de violences familiales ou conjugales dans son rapport de 2019, le défenseur des droits, déplore le fait que certaines préfectures continue de subordonner le renouvellement du titre de séjour ah, je cite : l'obligation de produire la preuve d'un divorce en cours, voire d'un divorce pour faute ou d'une condamnation pénale de l'auteur des violences, cette pratique ne tient pas compte de la réalité qui est celle des victimes des violences conjugales, elle n'est pas non plus conforme à la volonté exprimée par le législateur dans la loi de 2016 relative au droit des étrangers en France, en adoptant cette loi, le législateur a clairement entendu rendre automatique le renouvellement automatique le renouvellement du titre de séjour des étrangers victimes de violences conjugales ou familiales, malgré la fin de la communauté de vie j'ajoute que les juridictions administratives rappelle régulièrement que la preuve de violence peut être établie par tout moyen et que le renouvellement du titre de séjour n'est en tout état de cause, jamais subordonné à la condamnation pénale du conjoint violent. Alors cet amendement-là concerne donc 3 types de type de séjour, les cartes de séjour temporaires, vie privée, familiale, les cartes de résidents conjointe de Français après 3 ans de vie commune et les cartes de séjour temporaires regroupement regroupement familial, il vise à régler les conséquences d'une cessation de la vie commune pour violences conjugales en prévoyant un renouvellement de plein droit du titre de séjour permettant la preuve des violences conjugales, par tout moyen, toutefois, cet amendement est déjà satisfait, contrairement à l'autre, les bénéficiaires de ces types de séjours ne se font pas retirer leur titre du fait de la cessation de la vie commune et les textes en permettent déjà un renouvellement de plein droit, par ailleurs, en l'absence de précisions dans la loi, les faits de violence peuvent être trouvées par tout moyen, il est donc inutile d'apporter des précisions rédactionnelles suggéré qui risque de créer des interprétations à contrario peu favorable dans d'autres articles, il s'agit donc d'un problème de pratiques administratif qui peut être réglé par circulaire

vous le maintenez donc nous allons mettre aux voix, cet amendement, qui reçoit donc un un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Ces contres. S'abstient, il n'est pas s'adapter après l'article 12 bis, un amendement 62, il est présenté par Madame Lepage. Madame Lepage. Présidente la loi du 10 septembre 2018 a prévu la délivrance d'une carte de séjour aux seules victimes de violences conjugales, qui bénéficient d'une ordonnance de protection, or il est de fait notoire que très peu sont délivrés chaque année, nous avons déjà débattu du sujet plus tôt dans la journée afin de ne pas limiter la portée de cette mesure, le présent amendement prévoit de supprimer la condition de l'ordonnance de protection pour autoriser au séjour sur notre territoire, toutes les victimes de violences conjugales, si au terme des procédures judiciaires les faits de violence ne sont pas reconnus, il est prévu que la carte de séjour est immédiatement retiré. Chers collègues, avis de la commission madame la rapporteure. Sur le 62 merci madame la présidente, donc, cet amendement vise à assouplir les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en cas de violence conjugale ou de menaces de mariage forcé en l'état actuel du droit, ces violences ou une doivent être attestée par l'obtention d'une ordonnance de protection, les auteurs de l'amendement souhaite supprimer cette condition d'avoir obtenu une ordonnance de protection, arguant du fait que ces ordonnances sont trop difficilement accordés, ils apportent en complément, la précision que si, au terme des procédures judiciaires, des faits de violence ne sont pas reconnus alors la carte de séjour et immédiatement retiré, il semble toutefois vraiment souhaitable de s'en tenir au droit existant, la délivrance d'une ordonnance de protection et la garantie qu'un juge a apprécié la vraisemblance des faits et du temps chez encourus, ce qui évite tout détournement de ce fonds d'délivrance d'une carte de séjour temporaire, par ailleurs, contrairement à l'intention des auteurs de l'amendement si nous transfère l'appréciation au service de la préfecture, il n'est pas du tout certain qui se fonde sur une vraisemblance des faits allégués comme le prévoit le code civil en matière d'ordonnance de protection mais pourrait au contraire exiger une matérialité plus grande des faits, j'ajouterai que les ordonnances de protection sont désormais plus souvent délivrées par les JAF qui se sont dit qui se désole appropriée et que les étrangers s'en séjour régulier peuvent obtenir l'aide juridictionnelle, à ce titre, donc c'est un avis défavorable. Merci madame la rapporteure, Madame la Ministre. Même avis pour les mêmes motifs, la présidente. Même avis du Gouvernement je vous remercie, je mets donc aux voix l'amendement 62 avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Les contres. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, je mets aux voix, l'article 13 qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il est à 2. C'est après l'article 14 un amendement 19 il est présenté par Madame Benbassa. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État d'État, mes chers collègues, je souhaite ici attirer l'attention de notre haute assemblée sur des violences d'un genre nouveau, et encore largement méconnue, celle des violences administratives, celle-ci consiste pour le partenaire maltraitants à confisquer ou détruire les documents administratifs de sa conjointe ou compagne afin de la bloquer dans ses démarches et dans l'accès à ces droits ces pratiques entraîne une forme d'emprise de l'agresseur sur la victime qui se trouve totalement dépendante de son bon vouloir ces brutalités psychologique frappe particulièrement les personnes étrangères, les plaçant dans une situation de de grande vulnérabilité sur notre territoire pour ces personnes migrantes la rétention par leur conjoint ou compagnon de leurs documents d'identité de séjour ou encore bulletin de famille revient à avoir la peur permanente de ne pas pouvoir mener à bien certaines démarches administratives lourdes de conséquences, aux violences physiques et psychologiques pratiqués à leur endroit par leur agresseur s'ajoute ainsi la crainte de l'expulsion de la précarité sociale et financière cette emprise place la victime dans une situation de soumission et l'empêche d'acquérir une autonomie susceptibles de lui permettent de quitter son compagnon les souffrances verbale, psychologique, physique et sexuelle tendent aujourd'hui à être, il n'en est rien des violences administratives en raison de leur ignorance par les autorités. Ainsi est-il proposé par le présent amendement que dans les 6 mois suivant la promulgation de cette loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport à ce sujet, permettant ainsi au législateur de bénéficier de données chiffrées et documenté, afin que des solutions soient trouvées en la matière, je vous remercie. Si Madame Benbassa Madame la rapporteure, avis de la commission, merci, madame. Donc en fait il s'agit de d'une demande de rapport sur les violences administrative dans le cadre conjugal, donc plus qu'un rapport sur ces formes de violences, il convient de sensibiliser les pouvoirs publics à ces situations, et donc nous demanderons Madame la Garde des Sceaux, son voilà son regard là-dessus, donc c'est une demande de retrait concernant cet amour. Je vous remercie, madame la ministre à vie du gouvernement. Merci madame la présidente, madame la rapporteure, madame la sénatrice de. Alors je voudrais vous dire que je partage votre constat sur le fond, et d'ailleurs, ce sont des sujets qui sont beaucoup remontée du Grenelle des violences conjugales, notamment en ce qui concerne les moyens de paiement et le fait de subtiliser des moyens de paiement ou des papiers d'identité et c'est également un sujet qui nous a été remonté par les associations pendant la période de confinement des associations ont fait état de femmes auxquelles on a dérobé les attestations de sortie ou des stylos ou de quoi pouvoir écrire et donc sortir, donc je pense que ce que vous décrivez est tout à fait une réalité qui doit être mise au jour où débattu et c'est la raison pour laquelle nous avons créé un groupe de travail dans le cas du Grenelle des violences conjugales spécifiquement sur ce que nous avons appelée nous les violences économiques mais qui induit évidemment la question des violences administratives et je suis persuadé que ce groupe de travail parce que j'en ai réuni les pilotes, ce matin, sera tout à fait d'accord pour échanger avec vous, peut-être vous auditionner voir quel travail il est possible de faire au long terme pour avancer ensemble sur cette question, sur la base de de ce que vous proposez et je voudrais vous dire que je reçois jeudi l'ensemble des banques pour les mobiliser, les sensibiliser notamment sur en fait particulier qui nous est aussi beaucoup remonté, c'est-à-dire le moment où la femme souhaite quitter son conjoint et le conjoint, téléphone à la banque pour faire supprimer ces moyens de paiement, c'est une réalité qui nous a été rapporté à de nombreuses reprises, donc nous souhaitons les recevoir et je les reçois jeudi ou vendredi, afin de savoir quelles actions elle compte mettre en place pour mettre fin à cela qu'il est déjà interdit par la loi mais néanmoins qui se pratique encore, donc c'est une un avis défavorable du gouvernement pour le rapport en tant que telle, mais nous, nous enregistrons votre demande de mettre ce sujet à l'agenda et y travailler sérieusement. Si Madame la ministre madame Dumas ça vous maintenez votre amendement, nous mettons donc l'amendement voit avec donc une demande de retrait ou défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre. S'abstient, il n'est pas adopté après article le. 14 un amendement 58 rectifié de présenté par Madame Rossignol.

le soutien qu'apporte aux victimes et aux procédures, la présence intervenant social en gendarmerie en commissariat qui partout où ça existe sont salué comme étant un véritable accompagnement une aide à la fois d'ailleurs aux forces de police ou de gendarmerie comme aux victimes et en même temps, j'imagine qu'il vous aussi remonter le la situation de 16 départements qui sont en France dépourvue d'intervenants social en gendarmerie ou un commissariat cet amendement dans un monde idéal, c'est un monde où le Parlement aurait une large initiative de propositions dans les politiques publiques, nous aurions proposé que les dans les départements qui ou dans lesquels les les communes sont peu fortunés et dans lesquels aucun aucune collectivité locale ne s'engage suffisamment pour créer ces postes d'intervenants social nous aurions proposé que les communes puissent à 100 % financer ces intervenants sociaux je en en utilisant les fonds alloués par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, mais comme nous ne sommes pas dans un Mondial, nous ne sommes que dans le monde réel dans le monde réel, ce n'est qu'un amendement proposant un rapport sur le les la situation des 16 départements c'est un amendement qui a été à l'initiative de notre collègue Marie-Pierre Meunier, sénatrice de la Drôme et qui est cherche réellement auprès du gouvernement, l'appui nécessaire pour apporter aux victimes de la Drôme, le même appui que celui qui est apporté dans bien d'autres départements. Merci, cher collègue madame la rapporteure, avis de la commission.

si, on comprend, on est, on est d'accord avec le problème soulevé, mais bien qu'il soit caché, c'est quand même une demande de rapport et donc, nous appliquons la jurisprudence habituelle de la commission sur les demandes de rapport, nous ne sommes pas favorables au rapport, nous le disons régulièrement et avec beaucoup de constance aussi, mais nous sommes quand même bien favorable à l'accompagnement social des vies. Merci beaucoup madame la rapporteure, Madame la Ministre. Merci madame la présidence Madame la rapporteure, madame la sénatrice. L'augmentation du nombre de ces intervenants, a été, effectivement, vous l'avez rappelé prévu dans le cadre du Grenelle des violences conjugales et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, a fait savoir que 80 nouveaux postes était prévue sur l'année 2020 15 ont déjà été recrutés avant la crise liée à la pandémie de Covid 19 et comme l'ensemble des autres mesures du cadre du Grenelle des violences conjugales, cette mesure fait l'objet d'un suivi annuel dans le cadre d'un comité qui est composé de représentants de l'ensemble des administrations concernées du ministère de l'Intérieur, ministère de la justice, service des droits des femmes, direction générale de la cohésion sociale, etc et ces services seront appuyées d'un outil de report outil de report qui à tout moment par chacune des administrations poursuivre justement les implantations, territoire par territoire et ce comité, il est donc chargé de rendre chaque année en novembre dans la lignée des travaux conjoints entre l'administration en charge du suivi du Grenelle des violences conjugales, la DGCCRF et ses partenaires, incluant le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, un bilan précis de l'état d'avancement des mesures de graisse qui répond à la demande de rapport donc un avis défavorable. Merci madame la ministre, alors j'ai une demande d'explication de vote de Monsieur, la Mini. la présidente, madame le ministre, chers collègues, que le Comeau je dirais concernant cet amendement et serait que tous les amendements ont aussi un un bien-fondé, on le mérite aussi de poser aussi beaucoup de de problèmes et de préoccupation, même si cet amendement, c'est une demande de rapport, mais je me permettrais d'intervenir sur ce sujet-là, parce que, au sein de la délégation du droit des femmes, et tous les collègues la et la présidente Annick Billon c'est vrai que on on a souvent abordé ce sujet même, bien avant la crise sanitaire, on sait que la tâche est immense au sein des des interventions à caractère social qu'au fond les les policiers, les gendarmes même osciller les sapeurs-pompiers, enfin toutes les forces de sécurité civile, entre autres, qui interviennent aussi, et avant la Christine sanitaire, la situation était franchement franchement déjà pas simple, bon, après, avec cette crise sanitaire et et sous l'autorité des des représentants de l'État aux préfets, sous-préfets, vous savez, on avait quelques entretien téléphonique pour poser aussi c'est ces problèmes et avant la crise sanitaire, sous l'autorité des représentants de l'État, il y avait aussi le établir des bilans aussi à l'échelle des départements d'appartements, les Ardennes et on a la chance de voir des intervenants sociaux en gendarmerie ou police grand souci au partenariat avec les collectivités territoriales, conseil départemental, l'intercommunalité, voire comme mais se pose : d'un côté aussi ce problème de financement bien entendu tout et tout, et tout, et financier mais de l'autre côté il y a surtout le volet humain qui était largement mis en en évidence au fil je dirais de de l'examen de cette proposition de loi

le rapporteur, Madame la Ministre, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est c'est important vraiment et de et et et et de poursuivre : surtout, mais on sait que la tâche est immense et et on sait aussi qu'on peut compter sur l'ensemble des partenaires. monsieur Laménie je vais maintenant mettre aux voix l'amendement 58 rectifié, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. S'abstient, il n'est pas adopté après l'article 14 un amendement 59 rectifié, il est présenté par Madame Filleul. Madame Filleul. Présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, cet amendement est aussi une demande de rapport pour dresser un bilan des conséquences de la crise du coronavirus sur les violences conjugales reconnaissait cependant que les circonstances sont extraordinaires, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a été élaboré et voté à l'Assemblée nationale avant la crise sanitaire relative à l'épidémie de Covid 19 avant la période inédite de confinement qui a été un facteur aggravant des violences conjugales, pour autant, nous n'avons pas à ce jour de bilan sur l'ampleur de ce phénomène, nous savons cependant que la justice a tourné au ralenti et il y a un risque de voir les délais des audiences déjà important augmenter l'éventail des réponses pénales s'est réduit, les obligations de soins ont été renvoyés à la fin du confinement, tout comme celle de pointer au commissariat les stages de responsabilisation pour les auteurs normalement organisée par les services pénitentiaires d'insertion et de probation n'ont plus lieu, tout cela doit être mesurés afin de pouvoir éventuellement y remédier, nous devons pouvoir identifier les difficultés spécifiques qu'ont pu rencontrer ou que rencontrent encore les victimes de violences en raison du confinement, par ailleurs, si des mesures ont été prises par votre gouvernement, il nous faut pouvoir les évaluer évalue et éventuellement en tirer des enseignements, soit pour les améliorer, soit pour les pérenniser, si elles permettent de mieux lutter contre les violences faites aux femmes, nous devons également pouvoir identifier et analyser les manques ou les failles afin de pouvoir en tirer toutes les conséquences si cette situation était amenée à se reproduire. rapporteure. La présidente. Le confinement a été un épisode absolument inédit sans précédent, donc il est évident que l'impact du confinement sur les violences conjugales, très vite, on a su que ce serait identifié comme un enjeu de première importance, violences conjugales, violences sur les sur les mineurs, donc j'espère que que le gouvernement va pouvoir nous donner des éléments en séance des éléments chiffrés, des éléments détaillés, nous savons que vous aviez mis en place Madame dès son droit pour recueillir les plaintes que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit dans les pharmacies, nous savons aussi que l'Ordre des avocats avait ouvert une ligne gratuite de téléphone, donc j'espère que vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus et on aura besoin de ce bilan détaillé de ce bilan chiffré pour savoir vraiment ce qui s'est passé pendant ce ce confinement et donc à la lumière de ce que vous allez nous dire, nous pourrons répondre à notre collègue qui a rédigé cet amendement en attendant vous explications. Merci madame la rapporteure. Merci madame la présidente, madame la rapporteure, madame la sénatrice. Pour vous répondre d'abord dès la fin du mois de mars, j'ai confié une mission à Élisabeth Moir Umbro qui est magistrate, qui est secrétaire général de la Mission interministérielle de protection des femmes cette mission, elle consiste à lui demander de travailler sur l'évaluation de la prévalence des violences conjugales pendant le confinement et donc nous avons mis à sa disposition l'ensemble des indicateurs des administrations nécessaires à cela ce rapport cette mission, les résultats de cette mission seront rendues au mois de juillet et nous aurons donc à cet égard de manière indépendante par la magistrate Élisabeth Maurin. Une évaluation de la prévalence des violences conjugales, pourquoi, parce que on disait dans votre propos liminaire avec la garde des Sceaux, il y a davantage de signalements 5 fois plus de signalements sur la plateforme arrêtons les violences Point gouv Point FR 36 % d'appel aux forces de l'ordre, en plus, mais il y aurait, avec beaucoup de précautions, mais d'après les premiers résultats dont nous disposons, il y aura eu moins de féminicides, mais pour avoir de véritables résultats avec des indicateurs le plus précis possible j'ai confié cette mission à Élisabeth mon art Umbro qui va donc nous la remettre, par ailleurs, en ce qui concerne les dispositifs mis en place par le gouvernement, j'ai présenté il y a une quinzaine de jours publiquement les évaluations et les résultats chiffrés, donc ils sont à votre disposition sur, je crois, le site du ministère, en tout cas sur l'ensemble des réseaux sociaux et dans les médias puisque je l'avais fait à l'occasion d'une interview dans un média pour que justement tous ces résultats soient publiques donc nous pourrons vous les avez adressé, vous-même madame le rapporteur, madame la sénatrice et à tout parlementaire ou toute personne qui en fait la demande, puisqu'ils sont publics et que je les ai déjà présenté il y a une quinzaine de jours peut-être pour en rappeler brièvement certains il y a le dispositif d'alerte des forces de l'ordre dans les pharmacies qui a donné lieu à plusieurs gardes à vue à plusieurs comparution immédiate à plusieurs relogement d'hommes auteurs de violences conjugales dans plusieurs endroits du territoire, nous avons aussi ouvert avec le ministre de l'Intérieur, la possibilité de signaler les violences conjugales par SMS au 114 pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de téléphoner et nous avons eu énormément de de SMS qui ont été adressées au numéro du 114 nous avons également ouvert une ligne téléphonique avec la Fnac, la Fédération nationale d'autres d'accompagnement des auteurs de violences conjugales, pourquoi, parce que dans l'état d'esprit de ce que nous évoquions tout à l'heure, la prise en charge des auteurs de violences conjugales, nous avons considéré que pendant la période de confinement, il y avait peut-être des gens qui ne savaient pas gérer leurs accès de violence et qui avait besoin d'un accompagnement alors nous savons qui ça ne concerne pas tous les hommes, il y a des hommes violents qui prennent du plaisir à terroriser leur famille leur épouse, leur entourage, etc, il y a aussi des gens pour qui c'est une souffrance et qui ont besoin d'appeler et nous avons passé la barre des 500 appels depuis le début avril, où nous avons ouvert cette ligne téléphonique, donc à 500 reprises, un homme sur le point d'être violent a téléphoné a eu en accompagnement avec un psychologue, avec des experts et a pu avoir par exemple une une possibilité pour être logés, nous avons d'ailleurs également mis en place une plateforme de logement d'hébergement des auteurs de violences conjugales avec la garde des Sceaux et en partenariat avec le groupe SOS et ça nous a permis de reloger en moyenne en 3 heures les hommes auteurs de violences conjugales vs 48 heures en moyenne habituellement, d'après les magistrats, donc c'est un progrès et tous ces dispositifs, nous allons les pérenniser, de la même manière que les 90 points d'écoute et d'accompagnement des femmes que nous avons mis en place dans les hypermarchés et dans les centres commerciaux, rester ouvert grâce à l'engagement des associations locales de terrain pour lesquels nous avons débloqué davantage d'argent, c'est le fonds que j'évoquais tout à l'heure et pour terminer, je voudrais dire que ce confinement, il est arrivé, évidemment, de manière imprévisible en France mais aussi dans tous les autres pays, je suis en lien avec mes homologues en Italie, en Espagne, en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays et nous sommes en train de travailler avec l'administration aux droits des femmes, un plan de confinement pérenne qui permettra dans l'avenir, si d'aventure dans 6 mois, un an, 5 ans 20 ans la France devait connaître de nouveau une période de confinement, il y aurait à disposition ce plan de confinement déjà prêt avec l'administration pour les personnes qui seront à ce moment-là, en responsabilité, qui voudront le mettre en oeuvre sur la base de l'expérience malheureuse que nous venons de vivre, j'espère que cela répond à votre question.

Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Un moment donc à l'article 15 un amendement 20 rectifié Madame Benbassa c'est vous qui le présenter. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les violences conjugales, touche tous les pans de notre société, les couples de même sexe ne font hélas pas exception pourtant : nous ne sommes pas pour l'heure du mal renseignés sur l'ampleur de ce phénomène en effet la mission interministérielle pour la protection des personnes compte les violences qu'on conjugale ne communique des chiffres relatifs au aux victimes féminines sans faire mention du sexe de l'auteur de maltraitance, les seules données dont nous disposons à propos des brutalités au sein des couples de même sexe proviennent de l'association Agir qui a mené une étude en la matière, en 2013, selon ces chiffres, et 11 % des gays et des lesbiennes et 20 % des personnes bisexuelles déclare avoir subi des maltraitances conjugales, seulement 3 % d'entre elles ont alors porté plainte, ces éléments ne sont pas récents et manque de précision, faute de l'échantillon représentatif de la communauté LGBT dans sa globalité, il semble évident que toutes les violences conjugales ne saurait être traités avec les mêmes outils, l'action publique devrait donc être en mesure de s'adapter au profil de la victime ainsi est-il souhaité par le présent amendement que l'Arctique soit rétabli dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale afin que rapport puisse être remis au Parlement visant à rendent compte de la diversité des violences conjugales dans les couples de même sexe ce rapport permettrait d'adapter les dispositifs de plus de Charles, pardon, de prise en charge et d'accompagnement des victimes issues des couples homosexuels et lesbiens en tenant compte de leurs spécificités, je vous remercie. Si cher collègue, avis de la commission madame la rapporteure. La La présidente donc la commission vous savez et et par principe réservés sur les demandes de rapport, elle a donc supprimé la de rapports qui figurait donc à l'article 15 mais ça ne veut pas dire que le sujet qui était évoqué à l'occasion de cet amendement n'est pas intéressant, bien au contraire, la question mérite d'être abordé, mais est ce que nous avons réellement besoin d'un rapport au Parlement pour nous donner les moyens de mieux connaître le phénomène ou d'engager des actions de sensibilisation des professionnels concernés, on a un peu peur, je dois dire que les les rapports ça devienne un alibi pour ne rien faire. Merci madame la présidente, madame la rapporteure, madame la sénatrice. Alors, nous ne faisons pas rien sur cette question, je vais vous répondre d'abord nous avons accompagné le lancement d'une application qui est lancée par l'association Flag, une application que je marraine et que mon service finance en partie et qui permet justement de signaler à des policières et des policiers formés pour cela, les violences dans des couples de même sexe puisque l'association Flag regroupe des membres des forces de l'ordre, qui sont des personnes LGBT plus et qui sont donc engagés pour un meilleur accueil et une meilleure prise en compte de ces questions par ailleurs interpellé comme vous venez de le faire, madame la sénatrice par des associations de défense des personnes LGBT plus pendant le confinement qui disait : ce que vous dites, c'est-à-dire que, on ne connaît pas assez les chiffres et qu'on a besoin d'avoir davantage d'évaluation sur les violences conjugales dans les couples de même sexe, j'ai décidé d'ajouter un volet à la mission confiée à Élisabeth Morin que j'évoquais précédemment qui porte spécifiquement sur la question des violences conjugales pendant le confinement par les couples de même sexe et donc cela sera nous sera remis au mois de juillet par la magistrate Élisabeth et puis enfin, peut-être juste pour vous réponde sur la question des chiffres, j'entends souvent dire à ce que vous venez dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de chiffres, il n'y a pas assez donné, notamment sur les féminicides ou sur les morts violentes dans le couple, je rappelle que, depuis des années, je crois que ça fait peut-être 10 ou 15 ans et publié tous les ans par le ministère de l'Intérieur, l'étude dites études sur les morts violentes dans le couple, qui met en lumière à la fois les femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint mais aussi les hommes est également bien sûr les morts violentes dans les couples de même sexe nous vous rejoignons complètement sur le fait que c'est un tabou en double tabou qui doit être levé et que nous devons agir et les pouvoirs publics agissent, est ce que c'est par un rapport, c'était le choix de l'Assemblée nationale, le gouvernement donne un avis de de sagesse au Sénat sur ce rapport. Merci madame la ministre, je mets donc aux voix l'amendement. 20 rectifié, qui est pour. Qui est con. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Après l'article 15 un amendement 69 présenté par Madame Lepage. Merci madame la présidente, cet amendement vise à étendre l'article 21 de la loi de 2010 tiret 769 du 9 juillet 2010 qui prévoit une formation sur les violences intrafamiliales les violences faites aux femmes sur les mécanismes d'emprise psychologique ainsi que ça les modalités de leur signalement aux autorités administratives et judiciaires, cette extension vise spécifiquement les personnels des postes diplomatiques, en effet, les victimes de violences conjugales, qui réside à l'étranger sont souvent encore plus isolé que celles vivant sur notre territoire les ressources et personnes auxquelles elles peuvent s'adresser, peuvent être plus difficiles à identifier nos postes diplomatiques devraient pouvoir être un lieu où elles peuvent être informés quant à leurs droits, cet amendement prévoit donc une formation pour les agents consulaires afin d'accueillir au mieux ses victimes de violences conjugales. Si Madame la sénatrice, je donne la parole à Madame, la rapporteure. d'une formation sur les violences intrafamiliales les violences faites aux femmes sur les mécanismes d'emprise psychologique ainsi que sur les modalités de leur signalement aux autorités administratives et judiciaires, à l'instar de ce qui est prévu depuis 2010 pour d'autres fonctionnaires et des magistrats, les consulats ont déjà pour mission de conseiller les ressortissants français sur les démarches qu'ils doivent entreprendre vis-à-vis des autorités nationales, la formation devra donc nécessairement être adaptés à chaque contexte local et le mécanisme de sa mise en oeuvre, ainsi que de sa prise en charge ne paraissent pas évident, la question est cependant importantes, elle mérite d'être posée et je vous propose donc de demander l'avis du gouvernement. Merci madame la rapporteure, Madame le ministre. Merci madame la présidente, madame la rapporteure, madame la sénatrice. Nous, nous considérons que c'est une question évidemment éminemment important et qui doit être néanmoins nous ne sommes pas sur cela relève de la loi, puisque, à notre sens, la question de la formation des personnels dans des postes diplomatiques relèvent plutôt directement du programme de formation du ministère des Affaires étrangères, plus que d'un vecteur législatif et, plus globalement, nous tenons à rappeler que les questions relatives à la sensibilisation et à la formation sur les violences conjugales font l'objet du suivi que j'évoquais précédemment dans le cadre des comités de suivi des mesures du Grenelle des violences conjugales, donc pour nous ce serait plutôt un avis défavorable. Merci madame la ministre, je mets donc aux voix l'amendement 69 vous rangez donc à l'avis du gouvernement Madame la rapporteure, donc avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

Qui est contre. Il n'est pas adopté. Alors, après l'article 15 un amendement de rectifier, terre, il est présenté par Monsieur Régnard. Merci madame la présidente. Cet amendement prévoit que le rapport annuel de la situation des Français établis hors de France, remis par le gouvernement aux instances représentatives des Français à l'étranger fasse expressément mention des violences conjugales en y consacrant une nouvelle subdivision la détresse des Français à l'étranger victimes de violence qu'on juge, donc j'ai pu parfois être témoin, et d'autant plus grande qu'ils sont hors du territoire national, une détresse qui est accru par cet isolement de fête sans compter leur fragilité liée souvent à leur statut migratoire. Pourtant un sujet aussi grave, nous n'avons que très peu d'informations, l'objectif de l'amendement et donc d'obtenir des données chiffrées, ainsi qu'un suivi du sujet, tout en évitant la rédaction d'un nouveau rapport, une meilleure connaissance du sujet permettra une prise de conscience nécessaire à la mise en place d'un accompagnement plus des Français à l'étranger victimes de violences conjugales, je vous remercie. Merci, cher collègue Madame la rapporteure. Madame la présidente. Donc, en fait, chaque année, le ministère des Affaires étrangères, rend public un rapport sur la situation des Français établis hors de France, cet amendement propose que ce rapport comporte désormais des développements consacrés aux violences conjugales chez les Français de l'étranger comme ailleurs, donc l'idée est intéressante et je note que ce rapport comporte déjà des développements sur la sécurité des Français établis à l'étranger, les violences au sein du couple constitue un facteur majeur d'insécurité, il est donc légitime de consacrer des développements à cette question importante, c'est donc un avis favorable. Merci madame la rapporteure, Madame le Ministre, un avis de sagesse, merci madame la Ministre, et donc je mets aux voix Madame Lepage pour explication de vote. Je trouve la demande de Monsieur Régnard évidemment intéressante mais je trouve la réaction de la rapporteure, aussi bien que de la ministre étonnante, nous avions un collègue tout à l'heure, qui parlait de cohérence, je me demande où est la cohérence, on ne veut pas former les agents diplomatiques pour accueillir les Françaises en situation de violence et on on veut quand même avoir des statistiques là quelque chose qui m'échappe. Merci, cher collègue, madame la ministre, vous avez la parole. Merci madame la présidente, madame la sénatrice. Que les choses soient très claires, personne, je crois, et ici n'a dit qu'on ne voulait pas former les personnels diplomatiques, il s'agit de dire que ça ne relève pas de la loi, il y a énormément de choses comme vous savez très bien, qui sont faites et qui ne sont pas inscrites dans la loi, donc nous nous souhaitons évidemment qu'il y ait une formation et que l'on avance sur ces questions et d'ailleurs, l'engagement de Jean-Yves Le Drian, sur ces sujets et reconnue dans le monde entier, avec notamment des objectifs. Très important en matière d'égalité femmes-hommes et de diplomatie féministe que porte la France, nous sommes un des trois ou quatre fait dans le monde, a porté cette diplomatie féministe et d'ailleurs nous sommes reconnus par l'ONU, puisque nous allons pour cela accueillir en juillet 2021, le forum Génération égalité qui marque les 25 ans du Forum mondial de Pékin des droits des femmes, donc il ne s'agit évidemment pas de dire que nous n'allons pas former les personnels en poste diplomatique, il s'agit de dire que ça ne relève pas de la loi et que la en revanche, il s'agit d'un rapport annuel qui existent déjà, il s'agit de considérer que l'on peut faire un focus là non, je pense que ça serait peut-être plus de nature à vous réjouir, parce que ça veut dire que, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure on ne laisse pas tomber les personnes qui sont expatriés, au contraire, on considère que c'est un sujet d'importance qui mérite d'être mis à l'agenda. Si Madame la Ministre, alors je mets maintenant aux voix l'amendement de rectifier terre qui a reçu un avis favorable de la commission et une sagesse du gouvernement qui est pour. Les contres. Qui s'abstient, il est adopté, après l'article 15 un amendement 7 rectifié Monsieur Young. Merci madame la présidente, je je fais court, c'était une demande de rapport, mais je prends conscience qu'il existe déjà un rapport qui est celui que Monsieur Régnard a évoqué tout à l'heure, et donc je me rallie à son amendement. Donc vous retirer votre amendement, vous le retirer. Donc l'amendement 7 rectifié retiré, je vous remercie, après l'article. 15 un amendement 22 madame Lepage, vous le présenter. Les 4 amendements suivants 22 66 67 et 68 étaient des demandes de rapports sur des sujets différents, mais je les retire. Merci, cher collègue, et donc les amendements 22 66 67 68 sont retirés, nous passons après l'article 15 à l'amendement 83 il est présenté par Madame Cohen. Oui, donc c'est le dernier amendement, effectivement, il est question là dans la dans la dernière ligne droite de de beaucoup de de rapport, mais cette fois-ci je veux aborder une question concernant le protocole féminicides qui est mis en oeuvre en Seine-Saint-Denis ce dispositif expérimental est unique en France, prévoit que, suite à un féminicides, ou à une tentative d'une particulière gravité, le procureur de la République prend en urgence une ordonnance de placement provisoire des enfants, ceux-ci sont confiés au service de l'aide sociale à l'enfance pour évaluation et hospitalisée dans le service de pédiatrie Robert Ballanger pendant une durée de 3 à 8 jours, avec des droits de visite suspendues pendant cette durée, vous savez que 60 % nous l'avons dit des enfants qui sont témoins de violences conjugales, présentent des troubles de stress post-traumatique, en cas de féminicides, ce taux atteint 100 % et donc, afin de protéger les enfants et prévenir les troupes de comportement un partenariat original a été mis en place en 2014 dans les départements de Seine-Saint-Denis entre le Parquet du TGI de Bobigny, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis via l'Observatoire des violences envers les femmes et le service de l'aide sociale à l'enfance donc, une fois que ces enfants donc sont présentées dans le service de pied de pédiatrie une évaluation somatique et psychologique est effectué par les intervenants du service, tous formés à la victimologie le service de pédopsychiatrie se charge également d'assurer l'interface avec le tribunal, la police, les professionnels des services de protection de l'enfance, il garantit aussi le suivi de l'enfant après la sortie de l'hôpital soit en poursuivant les les soins parfois plusieurs années dans l'unité de psycho-trauma à l'hôpital Robert Ballanger soit en organisant le relais thérapeutique auprès d'une autre unité spécialisée cette expérience qui a fait ses preuves en matière de prise en charge thérapeutique des enfants ayant subi un tels traumatismes donc mériteraient d'être étendue à d'autres départements où le schéma départemental de l'aide aux victimes, a fait de la lutte contre les violences conjugales, une de ses priorités, c'est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement qui demande tout simplement au gouvernement de remettre au Parlement un rapport dans les 3 mois suivant la promulgation de cette loi sur la possibilité de généraliser le protocole en question, en fait, il s'agit d'un quelque part de, de voir que cette expérience est vraiment très positive et d'encourager à ce qu'elle soit pratiquée dans d'autres dans d'autres parties du territoire et c'est via donc cette demande de merci, Madame Cohen, la parole est à madame la rapporteure. mais, comme l'indiquent les auteurs de l'amendement, il est expérimental, donc, il faudrait donc qu'ils soient évaluées avant d'être généralisées et nous demandons donc au au gouvernement, quels sont les éléments dont il dispose sur l'évaluation, plutôt que de demander un rapport. Merci madame la rapporteure, madame la ministre. Adrien taquet, le secrétaire d'État chargée de la protection de l'enfance et avec d'autres membres du gouvernement, c'est à ça qu'a servi le Grenelle des violences conjugales notamment c'est-à-dire expérimenter ou plutôt relevé, pardon, les expérimentations sur le territoire qui sont des bonnes pratiques que nous pouvons généralisée et nous avons d'ailleurs commencé à le faire sur un certain nombre de choses qui faisaient partie de ce protocole féminicide il y a certains éléments que nous retrouvons d'ailleurs dans cette loi et dans les autres mesures du Grenelle des violences conjugales, je pense également, par exemple, la grille d'évaluation du danger qui est inspiré directement de travaux qui ont été menées en Seine-Saint-Denis ou à la roue des violences qui est également inspiré également des travaux qui ont été menées là-bas nous je voudrais pour conclure, vous dire que c'est un sujet qui est en train d'être travaillée par le groupe de travail du Grenelle des violences conjugales, consacrée aux violences intrafamiliales qui mélange différentes administrations sous le pilotage de la direction générale de la cohésion sociale et qui notamment a en son sein des personnes éminemment engagé en Seine-Saint-Denis, nous sommes plutôt défavorable au fait de produire un rapport qui ne viendrait que confirmer ce que vous venez de dire à madame la sénatrice en revanche nous sommes favorables au fait de poursuivre l'analyse de cette expérimentation et de voir comment, y compris en terme de moyens et en termes de partenariat avec les conseils départementaux avec les différentes collectivités, avec les différents acteurs sur place, il est possible d'étendre ce protocole. Madame la ministre, je à Madame Cohen. Oui, en fait, c'était le but de de de cet amendement, d'abord, c'était de faire connaître cette expérience à l'ensemble des collègues qui sont ici présents, simplement effectivement parce que j'ai, j'ai participé, comme d'autres sénateurs et sénatrices et parlementaires au rendu un du Grenelle et je pense que c'est effectivement important de pouvoir s'appuyer sur les bonnes pratiques, essayer de les élargir à d'autres territoires, donc à partir du moment où où c'est dans la le l'objectif en fait qui nous a été soumis ce soir je vais pas maintenir cet amendement, au contraire, je pense qu'il faut tout à fait soutenir cette démarche et espérer que ça soit élargie à d'autres territoires, donc je retire mon amendement. Merci Madame Cohen donc l'amendement 83 et retiré, et donc je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, y a-t-il des demandes d'explications de vote Madame Rossignol. en début de débat, nous allons voter cette proposition de loi les articles qui la composent, pour autant le la tâche reste grande devant nous et je déplore que bon nombre d'amendements que nous avons présenté n'ait pas été accepté par le gouvernement ou les ou mais est néanmoins été votées par le Sénat, ce qui est une bonne chose ou d'autres n'ont pas été voté par le Sénat ce texte n'auront pas avec la philosophie de la justice en matière de violence conjugale et je regrette qu'ils ne tiennent pas compte des 24 recommandations qui avaient été transmises à la garde des Sceaux, après les rapports d'inspection de l'inspection générale de la justice sur les homicides et surtout, ce texte ne rompt pas avec la philosophie, qui en fait voeu que en toutes circonstances, on cherche toujours à maintenir le lien avec le père que les droits des parents, les droits du père en l'espèce, porte toujours sur la protection de la mère et des enfants, et que on ne naît pas décidé d'encadrer davantage le travail des juges au regard de ce que nous évaluons aujourd'hui comme dysfonctionnement dans la protection des victimes de violences conjugales et d'homicides et féminicides voilà nous voterons ce texte nous n'avons pas l'impression d'avoir participé à une grande oeuvre législative, nous votons un texte, donc nous ne savons toujours pas qu'elles sont là, les moyens qui lui sont qui sont assorties une il y a toujours pas les moyens qui ont été demandées par les associations, donc c'est un moment de la vie parlementaire entre 2 textes probablement sur la lutte contre les féminicides.

madame la rapporteure chers Marie Mercier monsieur le président de la commission des lois et la commission des lois, qui a travaillé à améliorer le texte, qui arrivait de l'Assemblée nationale, remercié les ministres qui sont passés cet après-midi, avec qui nous avons pu débattre regretter comme ma collègue Laurence Rossignol, qu'un certain nombre et de nombreux amendements et en fait, n'aient pas réussi à convaincre notre hémicycle parce que finalement ils s'embrassaient, beaucoup de sujets et le texte embrasser déjà beaucoup de sujets donc l'inflation législative, qu'on a connu ces précédents moi va peut-être se poursuivent donc ça nous permettra probablement d'avoir ce débat parlementaire sur des sujets tels que la parentalité, l'inceste, la prostitution, des jeunes, la formation des acteurs, l'accompagnement des victimes, la sortie des parcours des agresseurs, la médiation, l'ordonnance de protection etc, les sujets ne manquent pas, mais en réalité, ce que je voudrais vous dire c'est que je pense qu'on poursuit tous les mêmes objectifs dans cette, dans cet hémicycle, et on ne réussira qu'ensemble, donc il faut véritablement qu'on partage l'objectif est qu'on partage les moyens d'y arriver et je pense qu'on arrivera à attendent ses objectifs à plusieurs conditions à condition un, de disposer d'un véritable arsenal législatif cohérent et complet à condition que les lois votées soient appliquées uniformément sur le territoire, donc ça ne sera pas uniquement des guides et des fiches pratiques qui feront que que on y arrivera, à condition que la volonté politique soit sincère et donc dotés de Budgets suffisants pour la mettre en application, donc travaillons tous ensemble pour que les conditions soient réunies afin de protéger les victimes de violences conjugales et j'assume, j'associe à mon propos, Dominique rien du groupe Union centriste qui était la chef de file pour ce texte. Merci, cher collègue, je donne la parole à Madame Cohen et puis ensuite pour conclure madame la rapporteure. Oui, moi j'ai j'ai trouvé comme chaque fois qu'on aborde les questions des droits des femmes et puis là, la question des, des, j'ai toujours, je trouve que le débat est toujours passionnant, il est passionnant, il voit les le, le, le chemin parcouru, il y a des évolutions et on voit aussi les résistances qu'il reste à à combattre, mais je regrette, comme je l'ai dit, au cours de, de, d'un amendement, je regrette qu'on aborde la question des violences faites aux femmes, par un certain, une succession de lois qui qui du coup sont tout à fait, parcellaires et vraiment je réitère la proposition que nous nous portons au niveau de de mon groupe, de faire en sorte qu'il y ait une loi cadre qui rassemble toutes les problématiques et qui traitent d'un même mouvement aussi tout un travail éducatif de prévention, d'accompagnement et puis évidemment ce que je veux dire aussi parce que il y a une prise de conscience très forte de la société du fait que les violences faites aux femmes sont systémiques que c'est un système, c'est le système patriarcal qui en est à l'origine, et que c'est c'est ce système qu'il faut combattre pour en débarrasser la société mais que ça passe effectivement par un budget conséquent que le travail qu'on peut faire ensemble avec nos différences, avec nos divergences au niveau de la haute assemblée ne doit pas apparaître comme un travail qui va porter des coups aux politiques publiques qui sont menées, mais, au contraire, qui cherche à les renforcer et notamment à soutenir le fait qu'il y a un budget digne de ce nom, qui soient accordés au ministère et je souhaite d'ailleurs que le secrétariat d'État devienne un véritable ministère dédié aux droits des femmes et qu'il y a un budget suffisant en termes financiers en termes humains et malheureusement, malgré les déclarations qui sont faites au plus haut niveau et c'est une bonne chose quand c'est le président de la République qui s'exprime sur ce sujet, mais on voit bien là que part compte au niveau des actes concrets, on n'est pas au rendez-vous de ses engagements, donc voilà ce que je, je regrette, alors on a fait un petit pas, nous aussi, nous allons voter cette loi, nous l'avions dit dès le départ et ma collègue, Esther Benbassa, qui paie, qui pilotait le texte pour nous la tout à fait affirmer également comme l'ensemble de mon groupe.

j'ai annoncé en discussion générale que mon groupe aller voter ce texte et et ce n'est pas pour pour le répéter mais pour me féliciter de la qualité des débats que nous avons eu ici depuis le travail en commission et Madame la rapporteure y est pour beaucoup, le Sénat a tenu son rôle de d'avoir enrichi ce texte, nous nous sommes loin d'épuiser tous les sujets qui ont été posées par ce texte, mais il n'y a pas si longtemps que ça, ce sujet des violences conjugales était allez on va dire négliger s'en préoccupe de plus en plus et il faudra certainement encore des propositions des lois et des projets de loi pour s'occuper sérieusement de de ce texte, cette proposition de loi est une Pierre comme une autre à l'édifice à cet édifice qui va prendre énormément de temps avant, avant d'aboutir, merci à tous ceux qui ont contribué, donc, à commencer par Madame, la rapporteure ici au Sénat bien évidemment aussi les membres du gouvernement. Si beaucoup je pense que je peux vous donner la parole madame la rapporteure pour conclure. Merci madame la présidente, mais Madame la Ministre, mes, mes chers collègues, je voudrais vous remercie vraiment pour ce travail collectif qui a permis quelques avancées et des avancées concernant l'ordonnance de protection concernant les dispositifs sur le bracelet anti-rapprochement et évidemment sur l'accès aux sites pornographiques des mineurs, c'était un un amendement, vous l'avez compris qu'il ne tenait beaucoup à coeur : l'amendement 92, alors pour vous dire que tout ce qu'on peut faire pour protéger les femmes et les enfants, faisons-le ensemble et que, finalement, là où il y a une volonté, on trouve le chemin merci. Merci beaucoup pour cette conclusion alors je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales et adopté, mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance mercredi 10 juin à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement, la séance est levée.